La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 20 juillet 2017 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. Conformément à l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, M. le président du Sénat a pris acte de la cessation, le vendredi 21 juillet, à minuit, du mandat sénatorial de Mme Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur, et de M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, par décret du 21 juin 2017 relatif à la composition du Gouvernement. Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, a fait connaître qu'en application de l'article LO 319 du code électoral Mme Noëlle Rauscent a remplacé, en qualité de sénatrice de l'Yonne, M. Jean Baptiste Lemoyne. Le mandat de notre collègue a débuté le 22 juillet 2017 à zéro heure. Au nom du Sénat, je lui souhaite la bienvenue parmi nous.

le siège de sénateur de Loir-et-Cher restera vacant jusqu'au prochain renouvellement de septembre.

semble important que le Sénat puisse recevoir les explications nécessaires. Or il n'y a pas de séance de questions d'actualité cette semaine et la séance des questions orales qui aura lieu demain portera sur des questions ayant précédé l'annonce de cette mesure.

d'après l'avenir déduit du passé », telle est l'équation, formulée par Auguste Comte, que nous devrons résoudre collectivement pour rénover durablement notre modèle social. Régler le présent », c'est trouver des solutions opérationnelles pour lutter efficacement contre le chômage de masse, qui frappe durement et frappe en premier lieu nos jeunes, nos seniors et nos travailleurs peu qualifiés, en particulier dans C'est aussi prévenir la précarisation et le mal-être au travail d'un nombre croissant d'actifs, en donnant plus de sens au travail lui-même. Pour ce faire, il convient de considérer l'entreprise comme une communauté humaine au service d'un objectif de croissance. C'est enfin permettre à nos entrepreneurs d'innover, de créer de l'emploi et de défendre avec audace et confiance l'excellence de la créativité et du savoir-faire français partout dans le monde, pour que notre croissance soit durable, inclusive et surtout riche en emplois. d'après l'avenir », c'est faire en sorte que les solutions soient pérennes et robustes face aux mutations de grande ampleur que nous pressentons déjà, qu'il s'agisse des révolutions technologiques, du défi écologique ou de l'accélération de l'internationalisation des échanges.

Déduit du passé », cela veut d'abord dire qu'il est indispensable de tirer les leçons de nos échecs collectifs de ces trente dernières années : échecs à changer le regard sur l'entreprise,

qui sous-tendent notre modèle social, à savoir celles de la République : l'égalité et la liberté, socles de la fraternité. Par conséquent, faire table rase du passé ou transposer un modèle étranger tel quel constituerait une erreur majeure. Rénover, c'est concilier ces trois temporalités : le présent, l'avenir et le passé. C'est donc adapter pour poursuivre, pour faire vivre en le rénovant un héritage auquel nous sommes attachés. Rénover le modèle social français, c'est faire en sorte qu'il produise davantage d'égalité et davantage de liberté dans le monde à venir. Cette ambition, empreinte de pragmatisme, a présidé à l'élaboration du premier texte de loi que j'ai l'honneur de porter, au nom du Gouvernement, devant la chambre haute cet après-midi. Ce texte constitue la première pierre d'un projet plus vaste de rénovation de notre modèle social, annoncé par le Président de la République pendant la campagne présidentielle, engagé par le Gouvernement et très attendu par nos concitoyens, comme en atteste l'issue des dernières échéances électorales. Le projet de loi d'habilitation pour le renforcement du dialogue social et les ordonnances qui en découleront n'ont pas la prétention de résoudre à eux seuls l'ensemble des défis que je viens de citer. de citer. Ils donneront leur pleine puissance en résonance avec les prochains chantiers que le Gouvernement engagera ces dix-huit prochains mois : réforme de l'assurance chômage et de la formation professionnelle, mais aussi réforme de l'apprentissage, que je défendrai conjointement avec le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et réforme des retraites, que portera la ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn. Ils s'articulent aussi avec l'action du Gouvernement en faveur de la diminution du coût du travail, de la baisse de la fiscalité et du soutien au pouvoir d'achat. me demanderez-vous, commencer par cette réforme plutôt que par les autres et pourquoi recourir aux ordonnances ? L'habilitation que nous vous demandons aujourd'hui pour cimenter cette première pierre est essentielle à l'équilibre global de la rénovation de notre édifice commun : le modèle social français. Sur la méthode, tout d'abord, je souligne que ce véhicule législatif n'est en aucun cas un blanc-seing, puisque c'est un mandat sur un champ et avec des objectifs

cette méthode nous offre l'opportunité d'expérimenter une démarche inédite de coconstruction simultanée, qui articule en permanence démocratie politique, d'où l'importance de nos débats cette semaine, et démocratie sociale avec les huit organisations représentatives des salariés et des employeurs. L'une ne peut aller sans l'autre si nous voulons aboutir à des solutions calibrées, opérationnelles, comprises par nos concitoyens, acceptées et dont la mise en oeuvre sera ainsi facilitée. J'en ai été encore plus convaincue convaincue par nos échanges en commission mardi dernier et par la première lecture à l'Assemblée nationale, ainsi que par les trois cycles de concertation approfondie avec les partenaires sociaux que nous venons d'achever. Nous faisons le diagnostic que notre droit du travail souffre de deux handicaps. D'abord, il est devenu peu à peu inadapté à l'économie de notre temps, non pas dans ses principes, mais dans ses détails les plus précis. Il a été

Tout texte législatif doit prendre en compte cette réalité. Ensuite, le droit du travail est parfois inadapté à la réalité de ce que vivent et de ce qu'attendent les entreprises, mais aussi les salariés. Il néglige trop souvent la capacité d'un employeur et de ses salariés à trouver le meilleur compromis à leur niveau, au bénéfice de leurs intérêts respectifs, voire de l'intérêt général.

Les salariés sont très demandeurs de ce type d'organisation du travail afin de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie privée. Aujourd'hui, il concerne 18 % des salariés et 61 % y aspirent. Le télétravail offre plus de souplesse, car il allège notamment le troisième temps, le temps de transport, toujours caché, mais très lourd au quotidien. Il favorise en outre le maintien de l'emploi dans les zones rurales.

les nouvelles formes d'organisation du travail liées au développement d'internet, il se trouve dans l'incapacité d'apporter, avec la réactivité et la sécurité nécessaires, des réponses pertinentes à ce bouleversement. Aujourd'hui, la demande est si forte que ni les salariés ni les entreprises ne sont sécurisés juridiquement dans un contexte de développement hors champ du télétravail, sans autre précaution que la condition du volontariat. Si le télétravail est un enjeu d'amélioration de la qualité de vie individuelle, il constitue également une formidable opportunité d'amélioration de notre qualité de vie collective et de maintien de l'activité sur nos territoires.

pour allier libération des énergies et justice sociale, et, en l'occurrence, pour répondre aux besoins de liberté et de sécurité à la fois des entreprises et des salariés. Alors, que proposons-nous ?

car nous croyons en la capacité des organisations syndicales et patronales comme en la capacité des employeurs et des salariés à apporter les solutions les plus pertinentes, au plus près du terrain, pour faire converger performance économique et justice sociale. Qui d'autre mieux qu'eux peut trouver le meilleur compromis en s'adaptant aux réalités quotidiennes ? quotidiennes ? Confiance dans l'avenir, car nous sommes déterminés à lever les incertitudes juridiques qui pèsent lourdement sur les relations de travail et brident l'embauche. Il n'y a pas de modèle social durable qui repose sur des règles inconstantes ou anxiogènes. égard, l'efficacité de la réforme passe par trois maîtres mots complémentaires et interdépendants, qui charpentent le projet de loi : subsidiarité, lisibilité, prévisibilité. Subsidiarité, car il faut impérativement mieux connecter la prise de décision à ceux qui devront la respecter. Dit autrement, nous voulons que les entreprises et les salariés puissent décider davantage des règles qui leur sont applicables et qu'ils soient coauteurs de la norme sociale. sociale. La majorité des règles, jusqu'au moindre détail, relève de la loi. D'apparence égalitaire, ce cadre normatif crée en réalité trop de rigidité, de formalisme et de complexité. Cela entame par essence la possibilité de les adapter à la vaste diversité des situations du monde économique et social. De fait, des droits justes inscrits dans le code du travail ne sont plus accessibles ; à cause

Pour ces quatre critères, le Gouvernement propose de libérer les entreprises de la partie inapplicable de l'obligation de déclaration en externalisant le contrôle de la situation des salariés par des examens médicaux. En outre, la prévention des risques chimiques doit faire l'objet d'une réflexion spécifique.

Un droit s'il est formel et inapplicable n'est pas un progrès. Pour être réel, le droit doit être exerçable, quelle que soit la situation ou la taille des entreprises. La complexité est trop souvent un obstacle à l'exercice de droits réels, pour les salariés comme pour les entreprises.

pour comprendre que, sans rien renier des droits fondamentaux fixés par la loi, nous devons desserrer l'étau de la norme trop détaillée et permettre aux entreprises et aux salariés de négocier les règles qui leur correspondent dans un cadre fixé par la loi.

indépendamment des attentes des salariés ou des particularismes des secteurs et des entreprises. Pourquoi ne pas laisser les entreprises et les représentants des salariés décider ensemble des priorités ?

Je tiens à le réaffirmer solennellement : la loi est et demeurera le cadre dans lequel la négociation de branche et d'entreprise se déploiera.

La loi doit définir l'essentiel, les principes, l'encadrement des acteurs, mais nous voulons décentraliser davantage la négociation opérationnelle pour trouver les meilleurs compromis de terrain, tout en garantissant le rôle de la loi en matière de droits fondamentaux, de droits fondamentaux, comme les droits à la formation et à l'assurance chômage, l'égalité entre les femmes et les hommes ou l'interdiction des discriminations ou du harcèlement. De la même manière, De la même manière, les règles fondamentales à la vie des entreprises, comme la nécessité d'avoir une représentation du personnel ou les normes de santé et de sécurité, ne seront évidemment La branche continuera de jouer un rôle important, et je dois d'ailleurs vous dire, comme je l'ai déjà fait devant la commission, qu'à la demande des partenaires sociaux, tant patronaux que syndicaux, nous avons finalement choisi de renforcer non seulement l'accord d'entreprise, mais également l'accord de branche, principalement pour tenir compte du très grand nombre de TPE-PME dans notre pays, lesquelles ont besoin de supports et de repères. Nous considérons que la clarification de cette articulation et la sécurisation de l'ensemble supposent de définir trois niveaux. Au premier niveau, les accords de branche priment impérativement sur les accords d'entreprise. C'est le cas pour les minima conventionnels, les classifications, la mutualisation des financements paritaires ou encore les compléments d'indemnités journalières. En outre, nous proposons d'ajouter aux accords de branche la gestion de la qualité de l'emploi : durée minimale du temps partiel et des compléments d'heure, régulations des contrats courts, conditions de recours aux contrats à durée indéterminée de chantier. d'une nouvelle capacité de négociation dans la branche. Bien évidemment, en l'absence d'accords de branche, c'est la loi actuelle qui continuera de s'appliquer. Notre système reste supplétif faute d'accord d'entreprise, c'est l'accord de branche qui s'applique ; faute d'accord de branche, c'est la loi, et, dans certains domaines, cela ne peut être d'ailleurs que la loi ou l'accord de branche. Autre point très important qui doit figurer dans tous les accords de branche : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

-les conditions et les moyens d'exercice d'un mandat syndical, la reconnaissance des compétences acquises et les évolutions de carrière des élus du personnel. C'est un point important. Si nous misons sur un dialogue social rénové, renforcé, plus proche du terrain, il faut que l'ensemble des acteurs soit en mesure de le mener.

C'est en permettant aux entreprises d'adapter leurs règles pour faire face, par exemple, à une hausse ou une baisse rapide de leur activité, en élargissant le champ de la négociation, en donnant plus de « grain à moudre » aux différents acteurs et en encadrant de façon pragmatique la liberté de négocier

Nous sommes l'un des rares pays à être dotés d'un système aussi complexe de représentation des salariés, puisqu'il existe quatre instances différentes dès lors que l'entreprise compte cinquante salariés. Outre son caractère chronophage pour les deux parties, cette segmentation prive les salariés et leurs représentants d'une vision stratégique

faut-il rendre plus lisible ce système, et simplifier et renforcer le dialogue social en réduisant le nombre de ses instances. Pour mettre fin à ce morcellement des négociations qui n'apporte rien aux uns et aux autres, nous proposons de fusionner les trois instances d'information et de consultation le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces trois instances formeraient une nouvelle entité que nous proposons d'appeler le comité social et économique. Par accord d'entreprise majoritaire ou de branche, ce comité pourrait aller plus loin et devenir une instance unique, dénommée conseil d'entreprise, intégrant également la compétence de négociation. évidemment pas de diminuer, à l'occasion de la fusion, le champ des responsabilités et des attributions des instances fusionnées. J'ai entendu les

fusionnée. Cette proposition ne vise en aucun cas à « baisser la garde » sur la santé et la sécurité au travail, sujets sur lesquels nous avons fait de très grands progrès collectifs ces dernières décennies.

Par ailleurs, pour obtenir un dialogue de qualité, il faut que les acteurs disposent des moyens appropriés. Le principe de recours à des expertises, que vous avez d'ailleurs encadré lors la discussion sur le nombre d'heures de délégation, la formation et les parcours de carrière font partie du sujet. C'est pourquoi j'ai confié à Jean-Dominique Simonpoli, directeur général de l'association Dialogues, une mission visant à recenser les pratiques les plus innovantes et avancées des branches et des entreprises en matière de parcours syndicaux, et à formuler des propositions opérationnelles dans ce sens. Celles-ci ont vocation à s'intégrer dans les ordonnances. Enfin, je sais que vous partagez avec moi le souci de trouver une solution opérationnelle pour encourager un dialogue social structuré, efficace et pragmatique dans les très petites et moyennes entreprises, qui, comme je l'ai déjà dit, constituent la majorité des entreprises et des salariés de notre pays. Ce n'est pas simple. L'intention est claire, mais il est vrai qu'après plusieurs décennies d'effort et l'adoption de nombreux textes on dénombre seulement 4 % de délégués syndicaux dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Le système actuel de mandatement ne fonctionne pas.

Les concertations sur ce sujet n'ont pas encore permis d'aboutir à une vision convergente. Nous continuons à y réfléchir, et je compte beaucoup sur nos débats,

L'insécurité juridique pénalise d'abord les entreprises, surtout les plus petites, qui ne connaissent pas parfaitement à l'avance les règles du jeu quand elles veulent se réorganiser, adapter leurs effectifs ou prendre des initiatives. L'enchevêtrement de normes peu lisibles doublé d'une jurisprudence évolutive et parfois inconstante est particulièrement dissuasif, d'une part, à l'embauche pour les petites entreprises et, d'autre part, pour les investisseurs étrangers. un tel arsenal normatif peut paraître protecteur pour les salariés, il est en fait souvent contre-productif, car les incertitudes et les rigidités qu'il génère conduisent non seulement à freiner l'embauche, notamment dans les petites entreprises, mais aussi à donner le sentiment que l'équité n'est pas au rendez-vous. La probabilité qu'un licenciement sur cinq se solde par un contentieux est une réalité. Les contentieux durent en moyenne 21,9 mois, et 29 mois en cas de formation de départage.

l'issue du contentieux devant les conseils de prud'hommes, pour le même préjudice et avec la même ancienneté, peut être très aléatoire : un salarié peut se voir octroyer des dommages et intérêts qui vont d'un à quatre en fonction du conseil devant lequel est portée l'affaire. Cela nuit à la à la prévisibilité et à la sécurité, ainsi qu'à l'équité. Les entreprises comme les salariés ont besoin de repères. C'est pourquoi nous voulons instaurer des barèmes planchers et plafonds pour les dommages et intérêts qui s'ajoutent aux indemnités de licenciement légales et conventionnelles. Une exception à la notion de plafond sera toutefois faite dans les cas de harcèlement et de discrimination, où il n'est pas seulement question d'emploi, mais aussi d'atteinte à l'intégrité de la personne. Il ne nous paraît donc pas pertinent de raisonner de la même façon. Plus largement, nous devons trouver un système qui favorise la résolution des litiges en amont en encourageant, lorsque la rupture est inévitable, la rupture conventionnelle, la transaction et la conciliation. Il ne s'agit donc évidemment pas de toucher aux indemnités de licenciement, qui sont connues à l'avance et clairement définies. J'ai d'ailleurs annoncé à l'Assemblée nationale l'engagement du Gouvernement à en augmenter le montant dans le même esprit de lisibilité en amont, préférable à une inflation du contentieux en aval. Restaurer un climat de confiance dans l'avenir en levant les incertitudes juridiques est indispensable pour assurer l'équité et la sécurité juridique tant des employeurs que des salariés, mais aussi et surtout pour restaurer la confiance dans une croissance porteuse d'emplois.

la difficulté à trouver les compétences requises. Il nous faut impérativement renforcer les compétences, à la fois pour répondre aux besoins des entreprises et pour doter les actifs de protections actives face au chômage. Pour cela, le levier de la réussite est la formation. C'est l'enjeu majeur du plan massif de développement des compétences des jeunes, des demandeurs d'emploi et de l'ensemble des actifs que le Gouvernement souhaite mettre en oeuvre dès cet automne sous la forme d'un plan d'investissement dans les compétences et, ultérieurement, de la réforme de la formation professionnelle que nous entendons mener. nous entendons mener. Nous sommes dans une situation paradoxale, avec des territoires où la croissance est repartie et où l'on ne trouve pas les compétences, et d'autres territoires où elle ne repart pas et où les demandeurs d'emploi n'ont pas d'espérance devant eux. L'investissement dans les compétences et la mobilité des actifs sont donc deux sujets essentiels. La réforme de la formation professionnelle s'inscrira dans le droit fil de l'existant tout en renforçant les droits individuels à la formation. Cette logique centrée sur l'individu doit aussi inspirer la réforme de l'assurance chômage,

Cette réforme y contribuera significativement, en induisant des changements profonds dans le sens d'une meilleure performance économique, d'une plus grande liberté, ainsi que d'une plus grande proximité et d'une décentralisation du dialogue social. Cette rénovation de notre modèle social a pour but de répondre non pas à des questions théoriques, mais aux vraies questions que se posent tous les jours les entreprises et les salariés quels qu'ils soient- ceux qui n'ont pas de travail et en voudraient, ceux dont la situation est précaire, les entreprises

par une réforme, qu'on annonce structurelle, de notre droit du travail. Il est indéniable que les employeurs, les salariés et ceux qui recherchent un emploi sont pénalisés par une réglementation trop rigide et parfois illisible, voire ubuesque. Le Sénat tente depuis plusieurs années d'apporter des solutions pragmatiques aux difficultés rencontrées par les acteurs économiques sans remettre en cause les droits fondamentaux des salariés. Le Gouvernement semble partager notre volonté d'adapter notre modèle social aux réalités de l'économie du XXIsiècle. C'est pourquoi nous approuvons la philosophie du présent projet de loi d'habilitation. ce soutien n'est pas inconditionnel, madame la ministre. Des sujets essentiels aux yeux de la majorité sénatoriale, comme la fixation par accord de la durée hebdomadaire du travail ou le relèvement des seuils sociaux, sont absents du texte. Le risque d'alimenter par ordonnances l'inflation législative, que dénonce avec raison le Conseil d'État, ne doit pas non plus être sous-estimé. Quant à la méthode retenue, elle est pour le moins singulière et sans précédent depuis 2007. Certes, il n'y a pas de recette miracle pour réformer le code du travail. Le précédent gouvernement avait d'abord privilégié la négociation d'accords nationaux interprofessionnels, avant de prendre la responsabilité de réformes législatives. Mais il s'est arrêté à des demi-mesures sur lesquelles sa majorité s'est déchirée et qui n'ont pas véritablement traité les problèmes de fond Le nouveau gouvernement a, quant à lui, décidé d'agir sans tarder, dès le début du quinquennat. Il y a effectivement urgence. Trop de temps a été perdu. Des discussions ont été menées simultanément au Parlement et avec les partenaires sociaux sur près d'une quarantaine de sujets techniques, mais d'inégale importance. Les orientations du Gouvernement demeurent toutefois floues changeantes, pouvant tout aussi bien témoigner d'une stratégie réfléchie que d'une succession d'hésitations. Nous ignorons à ce jour quelle sera la portée réelle des futures réformes. Madame la ministre, nous pouvons parfaitement comprendre que, sur certains sujets, vous nous demandiez une habilitation de principe, vous laissant le temps de la concertation et de la réflexion. Je pense, par exemple, à l'articulation entre accords de branche et accords d'entreprise, question à laquelle il n'y a pas de réponse évidente. En revanche, sur d'autres points que vous avez prévu de trancher rapidement, avant la fin de l'été, nous aurions parfaitement pu débattre dans le cadre d'un projet de loi ordinaire. Vous avez d'ailleurs relevé, devant la commission, que le Sénat avait pu se forger une idée très précise des enjeux en cause lors des discussions de différents textes ces dernières années. Comment encourager les accords collectifs dans les petites entreprises ? Quel régime appliquer au licenciement d'un salarié qui refuse un accord ? Quelles compétences donner à l'instance unique ? Quel délai raisonnable prévoir pour contester un licenciement ? Quel périmètre géographique retenir pour apprécier les difficultés économiques d'une entreprise appartenant à un groupe ? lors de la discussion des projets de loi Rebsamen, Macron et El Khomri. Nous connaissons les positions des différentes organisations représentatives et nous savons qu'elles ne sont pas d'accord entre elles, mais c'est notre responsabilité de législateur d'apporter des réponses claires. Et c'est parce qu'elle a pris ses responsabilités que la commission des affaires sociales a précisé les habilitations demandées, même si elle n'est pas opposée à ce que la rédaction détaillée des différents textes nécessaires soit déléguée à l'exécutif sous la forme d'ordonnances. Nous n'accepterons donc pas que l'on nous reproche d'avoir préjugé de l'issue des concertations. Celles-ci se sont d'ailleurs achevées vendredi dernier.

C'est pourquoi la commission des affaires sociales a adopté une trentaine d'amendements visant à renforcer l'ambition du projet de loi autour de trois objectifs développer la compétitivité et l'attractivité de l'économie, tenir compte des spécificités des petites entreprises et rationaliser notre droit du travail au profit des salariés et des employeurs.

en leur absence, directement avec le personnel, sans interdire, bien entendu, le recours au mandatement. Nous souhaitons ainsi développer le dialogue social dans les petites entreprises en valorisant le rôle des délégués du personnel. La commission soutient la volonté du Gouvernement d'encourager les référendums en entreprise pour valider un accord, mais l'employeur doit pouvoir en prendre l'initiative, et pas uniquement les syndicats. obligé les signataires d'un accord de branche à accorder une attention particulière aux petites entreprises dépourvues de représentants du personnel. du licenciement des salariés refusant l'application d'un accord collectif, nous avons tranché en faveur d'un motif spécifique afin d'unifier les régimes actuels. Nous avons écarté l'application des règles du licenciement collectif à ces salariés, tout en invitant le Gouvernement à les faire bénéficier d'un dispositif d'accompagnement équivalant au contrat de sécurisation professionnelle. La commission est revenue sur la disposition adoptée par l'Assemblée nationale qui réduisait de trois ans à dix-huit mois le délai prévu pour la restructuration des branches. Elle a refusé d'accélérer la généralisation des accords majoritaires en raison du blocage du dialogue social qu'elle pourrait entraîner. À l'article 2, nous avons approuvé la fusion des institutions représentatives du personnel en une instance unique et lui avons donné compétence en matière de négociation des accords d'entreprise, sauf accord majoritaire contraire. Nous avons souhaité que l'ordonnance traite de la formation des membres de cette nouvelle instance, sujet crucial en raison de l'étendue de ses missions. Le nombre de mandats successifs de ses membres a été limité à afin de garantir un lien entre les élus et l'activité quotidienne de l'entreprise. Les obligations en matière de transparence financière applicables aux comités d'entreprise, qui ont vu le jour grâce à la pugnacité de notre collègue Catherine Procaccia, devront par ailleurs être étendues à l'instance unique. Enfin, tout recours à une expertise devra être précédé d'une mise en concurrence pour limiter les coûts supportés par les employeurs. Soucieuse de lutter contre l'instabilité du droit, la commission a en outre supprimé trois demandes d'habilitation. La première, à la rédaction imprécise, visait à augmenter le nombre de sujets soumis à un avis conforme des institutions représentatives du personnel, au risque de remettre en cause le pouvoir de direction de l'employeur. prévoyait de modifier la représentation des salariés dans les conseils d'administration des grandes entreprises, alors même qu'aucune évaluation des dispositifs mis en place depuis 2013 n'a été réalisée et que la dernière réforme date seulement de 2015. Quant à la dernière habilitation, elle autorisait une refonte des missions des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, les CPRI, qui n'ont été installées que le 1 juillet dernier et auxquelles le Sénat s'est toujours opposé. À l'article 3, la commission a autorisé l'employeur à rectifier dans la lettre de licenciement les irrégularités de motivation sans incidence sur la cause réelle et sérieuse du licenciement. Nous avons souhaité la réduction au moins de moitié du délai de contestation d'un licenciement économique, actuellement fixé à un an. Nous avons également adopté un amendement ayant pour objet d'ouvrir un débat sur le coût des inaptitudes d'origine non professionnelle qui pénalisent parfois fortement les petites entreprises. À l'instar d'un grand nombre de nos voisins européens, nous avons retenu un périmètre national pour apprécier la cause économique d'un licenciement collectif lorsqu'une entreprise appartient à un groupe international. Ce faisant, nous avons souhaité combler un vide juridique qui permet au juge de choisir un périmètre européen, voire mondial, pour contrôler le bien-fondé d'un licenciement économique nuisant gravement à l'attractivité de notre territoire. Enfin, nous avons précisé que les accords de branche fixant les règles d'utilisation du CDI de chantier devront respecter un cadre fixé par la loi afin de garantir un socle commun aux salariés et aux employeurs relevant d'une même branche.

je rappellerai que l'une des causes de l'abandon de la réforme en 1973 était l'effet psychologique du « bas de la feuille de paie » et la crainte d'une détérioration des relations entre employeurs et salariés. Sans doute le même écueil guette-t-il la réforme du prélèvement à la source votée en décembre dernier. Par ailleurs, si le dispositif inscrit à l'article 60 de la loi de finances pour 2017 est sans doute l'un des projets les plus aboutis d'instauration du prélèvement à la source en France, il s'illustre aussi par son extrême complexité et ses imperfections.

Elle instaure en effet un système d'impôt sur le revenu à deux étages, dans lequel de nouvelles règles d'assiette et de taux propres au prélèvement à la source viennent s'ajouter aux règles actuelles de calcul de l'impôt. De plus, De plus, le prélèvement à la source présente des inconvénients notables pour les contribuables, comme l'absence de prise en compte des réductions et crédits d'impôt dans le montant du prélèvement, ou encore des conditions de recours au taux « neutre » particulièrement dissuasives

L'étude commandée par la délégation aux entreprises du Sénat qui nous a été présentée récemment confirme, quant à elle, les coûts d'adaptation élevés inhérents à la collecte de la retenue à la source par les entreprises. Au total, ce coût est estimé à 1,2 milliard 1,2 milliard d'euros, dont les trois quarts pèseraient sur les très petites entreprises. Dans cet article 9, le Gouvernement justifie le report d'un an par la nécessité d'« assurer un meilleur accompagnement dans la mise en oeuvre de la réforme » et d'approfondir les travaux de préparation. Il faut croire que tout n'était pas si prêt

En dépit des efforts importants fournis par les services de la direction générale des finances publiques, la fiabilité du dispositif est encore incertaine. En complément de l'expérimentation qui sera menée cet été avec les entreprises et les collectivités territoriales volontaires, qui ne sont d'ailleurs pas très nombreuses, le Gouvernement propose ainsi de réaliser un audit concernant la « robustesse » de la réforme et la charge induite pour les tiers collecteurs. Il eût certainement été préférable de faire figurer cette mesure de report dans un autre texte que le présent projet de loi d'habilitation, qui renvoie à un tout autre débat que celui du prélèvement à la source. Toutefois, une intervention rapide est sans doute nécessaire pour clarifier le traitement des revenus perçus par les contribuables en 2017 et éviter que leur taux de retenue à la source ne soit transmis aux employeurs à l'automne prochain. Dans l'attente des résultats de l'expérimentation et de l'audit mené par le Gouvernement, il serait prématuré de supprimer le prélèvement à la source. Pour autant, je souhaite non pas, et c'est d'ailleurs la position très majoritaire de la commission des finances, que nous en restions au, mais que nous recherchions

et contemporain, c'est-à-dire sur la base des revenus présents, de l'impôt sur le revenu. Ce dispositif reposerait sur un système d'acomptes, dont le montant pourrait être modulé à tout moment par le contribuable en cas de variation des revenus ou de modification de sa situation familiale. C'est tout le sens de l'amendement que nous avons adopté et dont l'objet est d'enrichir le contenu du rapport qui devra être remis par le Gouvernement au Parlement avant le 30 septembre prochain. Nous pourrons ainsi disposer de toutes les informations utiles avant de statuer sur l'avenir du prélèvement à la source. Remettons donc le débat de fond, et réjouissons-nous de ce report

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce projet de loi d'habilitation constitue une nouvelle agression contre le droit du travail, qui-faut-il le rappeler ?-organise la protection des salariés face à la puissance patronale et à celle de l'argent. Le code du travail n'est pas un frein au développement de notre société ; il est le fruit de décennies de luttes sociales pour imposer l'humanisme face à la dictature du profit. Le code du travail, c'est l'expression de la spécificité française

expression du peuple souverain, qui a longtemps garanti les droits fondamentaux des salariés. En toute logique, le projet de loi que nous examinons remet en cause tout ce qui constituait le programme du Conseil national de la Résistance : suppression de l'assurance chômage, suppression du régime de retraites par répartition ... Dans les ordonnances, antidémocratiques par essence, vous avez l'intention de fusionner les quatre instances représentatives du personnel, de plafonner le niveau des indemnités prud'homales en cas de licenciement, d'étendre la primauté des accords d'entreprises sur les accords de branches et de généraliser le recours aux CDI de chantier. Vous poursuivez la démolition pure et simple du code du travail. Ce faisant, c'est l'ensemble du pacte républicain issu de la Résistance que vous déstabilisez. La loi, vous la voulez pour servir l'économie et non plus pour satisfaire les besoins humains et sociaux. Elle devient un outil de dérégulation, alors même que les constituants de 1946 et de 1958 l'ont élaborée comme une protection des plus faibles. faibles. Qu'importe le stress au travail, les cadences infernales, les suicides sur les lieux de travail ! Leur diminution et leur suppression, ce n'est pas votre priorité Ce qui importe, c'est de répondre encore et encore au du profit, qui exige toujours plus de disponibilité, de compétitivité et de rentabilité et donc toujours plus de précarité pour les travailleurs L'État est censé garantir les droits des travailleurs énoncés dans le Préambule de la Constitution de 1946 face à la loi du marché. Les sénatrices et les sénateurs communistes considèrent qu'il importe, pour des raisons sociales, économiques, environnementales, de faire prévaloir le social sur l'économie. Cette conception d'une économie au service des hommes, qui se construit par solidarité et non par la concurrence, nous la nommons « société de progrès ». Les exigences d'un nouveau monde sont celles de la construction d'une société de partage et de solidarité, d'une société qui protège les droits et les développe. Tel était le sens du Préambule de la Constitution de 1946. Vous devez cesser cet affichage trompeur de la modernité, alors que vous faites ressortir les vieilles ficelles libérales. Nos concitoyens commencent à voir clair dans votre jeu- un jeu libéral

les salariés seront contraints de négocier individuellement non seulement leur contrat de travail, mais aussi l'ensemble des droits qui ne seront plus couverts par les accords de branche. Nous sommes là au coeur de votre projet : l'individualisation de la négociation, de l'organisation et de la durée du travail, voire de leurs droits à la protection sociale ! Avec vous, c'en est fini de notre société de solidarité et d'égalité ! Ainsi, de manière insidieuse, vous répondez à une demande ancienne et récurrente du patronat et du MEDEF, laquelle consiste à mettre fin à toute conception collective du travail pour renvoyer la relation de travail à la seule relation individuelle entre employeurs et salariés, que vous dénommez désormais collaborateurs ou associés. Vous tentez, par exemple, de faire croire aux salariés qu'il est possible de se libérer en devenant son propre patron. Sauf que cet eldorado n'est pas aussi rose que vous voulez le faire croire ! En 2016,

82 000 euros pour la vente et 32 900 euros pour la prestation de services. De fait, les trois quarts des entrepreneurs toujours actifs après trois ans déclarent un chiffre d'affaires inférieur à 15 000 euros par an

il est indispensable de garantir aux travailleurs la possibilité de se syndiquer et d'avoir recours à des représentants syndicaux pour défendre leurs droits. Le sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 garantit que « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Ce principe est remis en cause dès lors que l'on individualise les relations entre les travailleurs et l'employeur, qui peut organiser un référendum dans l'entreprise pour faire accepter les baisses de salaires. Il est tout de même contradictoire d'annoncer vouloir renforcer le dialogue social et d'utiliser, dans le même temps, tous les moyens possibles pour marginaliser les organisations syndicales dans les entreprises, par exemple, en fusionnant les instances représentatives du personnel ou en cassant le monopole syndical. Personne n'ignore que le syndicalisme se construit précisément sur l'exigence de la défense collective d'intérêts collectifs. Votre texte est, ensuite, contraire à la décision du 28 décembre 2006 du Conseil constitutionnel, qui garantit le droit des travailleurs à participer à la détermination collective des conditions de travail. Ce droit n'est plus effectif dès lors que le comité d'entreprise, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le délégué du personnel et le délégué syndical sont fusionnés en une seule instance.

L'instance unique aura-t-elle la personnalité juridique ? Pourra-t-elle ester en justice ? Madame la ministre, vous aviez pourtant participé à la rédaction d'un rapport sur la santé et le bien-être au travail, lequel préconisait « la mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental interentreprises pour prendre en charge les risques psychosociaux au sein des petites entreprises ». vous décidez de faire disparaître totalement les CHSCT ! En supprimant le CHSCT, vous remettez en cause l'action des syndicats pour que soit enfin reconnue l'importance des règles de protection de la santé

Cette instance unique va encore éloigner les représentants du personnel des salariés. Il s'agit clairement d'une entorse au droit des salariés à participer à la gestion de leur entreprise, droit garanti par le huitième alinéa du Préambule de 1946. Vous remettez en cause le monopole syndical en matière de négociation dans les TPE-PME. Vous ouvrez la porte à des élus du personnel sans indépendance vis-à-vis du pouvoir patronal et à des négociateurs subordonnés à la direction de l'entreprise. Mais il y a plus ! Outre l'individualisation, avec ce projet de loi, vous inversez également la hiérarchie des normes en étendant le champ de la primauté de l'accord d'entreprise. Vous faites la

Ne tentez pas de nous faire croire que les salariés auront quoi que ce soit à gagner dans cette concurrence entre entreprises. Le marché du travail est tel que ce ne sont plus les salariés qui font valoir leurs droits : ce sont les employeurs qui imposent leurs exigences. Le patronat parviendra toujours à s'organiser pour proposer le moins-disant le plus défavorable aux salariés. Quand il s'agit de gros sous, on peut leur faire confiance ! ( Les grands magasins vont pouvoir faire du chantage à l'emploi en demandant la réduction de la plage horaire du travail de nuit : la tranche de vingt et une heures à six heures pourra être raccourcie demain pour répondre aux désirs des acheteurs nocturnes impulsifs ! Enfin, votre texte porte atteinte à la justice prud'homale en plafonnant les indemnités en cas de licenciement abusif. Initialement prévue par la loi Macron et censurée par le Conseil constitutionnel, la loi El Khomri avait repris cette mesure ne soit retirée face à la mobilisation sociale. Pourquoi insistez-vous donc tant pour limiter le montant des dommages et intérêts versés au salarié ? Parce que ce plafond imposé aux juges prud'homaux sera une provision comptable pour les entreprises qui souhaitent licencier librement ! L'employeur pourra ainsi choisir de respecter le droit du travail ou prendre le risque d'une condamnation, car il connaîtra à l'avance le montant de l'indemnité. Côté salarié, c'est le règne de l'arbitraire Le projet de loi d'habilitation est ainsi contraire à l'article XVI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 garantissant le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, ainsi que le respect d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties. L'équilibre des parties est rompu dès lors que l'employeur peut donner le motif de licenciement. Le patron pourra ainsi évoquer le motif de son choix pour éviter un licenciement sans cause réelle et sérieuse. réelle et sérieuse. Robespierre, le 10 mai 1793, proclamait ... Où va-t-on ? ... que, « jusqu'ici, l'art de gouverner n'a été que l'art de dépouiller et d'asservir le grand nombre au profit du petit nombre et la législation le moyen de réduire ces attentats en système. Les rois et les aristocrates ont très bien fait leur métier. C'est à vous maintenant de faire le vôtre, c'est-à-dire de rendre les hommes heureux et libres par la loi ». Veuillez conclure, madame Assassi. Votre projet, madame la ministre, est un retour à l'ancien monde, celui de l'oppression par les puissants ! Il est contraire à la République sociale, à notre Constitution et à ses préambules. Il est un acte de régression lourd de conséquences pour notre peuple. Telles sont les raisons qui ont poussé mon groupe à déposer cette motion d'irrecevabilité. La parole est à M. Yves Daudigny, Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le groupe communiste républicain et citoyen, au travers de cette motion, nous invite à nous interroger sur la recevabilité du projet de loi.

Je n'utiliserai pas d'arguments autres que juridiques pour répondre à une argumentation qui est juridique. Je ne m'appesantis pas sur le second moyen soulevé, relatif à la méconnaissance de règles législatives, dès lors qu'elles n'ont, par définition, aucune valeur constitutionnelle. Elles n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article 44, alinéa 2, du règlement du Sénat. S'agissant de la méconnaissance du Préambule de la Constitution de 1946, je peine à trouver les articles auxquels vous faites allusion. Vous avez mal cherché ! Le droit de travailler et d'obtenir un emploi Le droit de défendre ses intérêts par l'action syndicale ? Le droit à la détermination collective des conditions de travail, ainsi qu'à la gestion des entreprises par l'intermédiaire des délégués ? Le droit de grève peut-être Au-delà d'une approximation de la base légale qui fonde la motion, je ne vois, dans le Préambule de 1946, que des articles qui viennent en soutien des objectifs fixés par le projet de loi d'habilitation- soutien de l'habilitation et non, aujourd'hui, de la ratification. Le champ de l'habilitation du présent projet de loi vise, en particulier, à favoriser le dialogue social. Il encourage employeurs et salariés à trouver le meilleur compromis à leur niveau, au bénéfice de leurs intérêts respectifs. Il ne me semble pas que le Préambule de 1946 y fasse obstacle.

Ces quelques considérations conduisent à conclure non seulement que le projet de loi n'est pas contraire au Préambule de la Constitution de 1946, mais aussi qu'un texte est certainement nécessaire pour poursuivre la réflexion sur l'évolution du droit du travail engagée lors du précédent quinquennat. L'avis défavorable que j'émets à l'égard de cette motion ne présage bien sûr en rien l'issue des votes sur le projet de loi d'habilitation et encore moins sur le futur projet de loi de ratification. Il est avant tout question d'ouvrir le débat. L'adoption de cette motion priverait le Sénat d'une discussion utile. Elle priverait l'ensemble des sénatrices et des sénateurs d'une tribune. Elle nous priverait surtout d'un examen complet du projet de loi en séance publique. Mes chers collègues, je vous invite, au contraire, à faire vivre la démocratie parlementaire et le bicamérisme ! Quel

tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité. Je ne partage évidemment pas leur analyse. Je me limiterai à trois exemples emblématiques. Premier exemple, l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que « tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». Ce principe constitutionnel ne fait pas obstacle à ce que le législateur distribue les compétences entre l'accord de branche et l'accord d'entreprise, comme l'a reconnu le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 avril 2004 sur la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. Une seule limite est posée : la loi doit fixer les dispositions d'ordre public. Le Gouvernement est donc fondé à rationaliser, à l'article 1, l'articulation entre accords de branche et accords d'entreprise. Deuxième Deuxième exemple, l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 prévoit que « tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. » Je précise qu'aucune disposition du texte ne remet en cause ce principe. La commission a souhaité renforcer le dialogue social dans les petites entreprises dépourvues de délégué syndical, mais tout salarié demeure, bien d'être désigné délégué syndical et l'employeur pourra toujours conclure un accord avec un salarié mandaté. Troisième exemple, le Conseil constitutionnel a considéré, dans sa décision du 5 août 2015, que le principe même

vote. Jusqu'à présent, je croyais que les syndicats et les communistes défendaient les salariés. Je constate qu'il n'en est rien

au début de l'année 2018, soit à peine quelques mois après la date de publication prévue pour vos ordonnances. Force est de constater que vous ne donnez pas l'impression de rendre ne serait-ce qu'à votre majorité parlementaire par extension, au Parlement tout entier la confiance qui vous a été donnée. Cela, vous me l'accorderez, va à l'encontre du renforcement du dialogue. C'est d'autant plus regrettable que nous aurions pu nous retrouver sur certains objectifs, par exemple, sur l'ouverture des droits à l'assurance chômage pour les salariés démissionnaires ou les indépendants. Au-delà du peu de confiance que vous accordez aux parlementaires, je tenais donc, madame la ministre, à vous rappeler que ces ordonnances feraient suite à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui a mis en place de réelles contreparties progressistes

Vous proposez cependant d'aller d'ores et déjà beaucoup plus loin dans le sens d'une restriction drastique de la régulation nationale au profit du moins-disant social avec, pour seul lot de consolation, le droit de discuter dans l'entreprise sur deux ou trois points qui seront listés par vos soins.

de loi, nous contestons le choix des ordonnances. Nous sommes sur un champ législatif très large, aussi vaste et complexe que le code du travail, et, en quelques jours de débat parlementaire, nous devrions valider le cadre que vous nous proposez, sans connaître tout ce qui s'est dit avec les organisations représentatives. Tout cela s'apparente à un blanc-seing ! Je rappellerai donc aux sénatrices et sénateurs qui s'apprêtent à vous suivre qu'ils abdiqueraient encore un peu plus leur pouvoir constitutionnel d'élaboration de la loi. En effet, même si, au final, les ordonnances n'étaient pas ratifiées par le Parlement, celles-ci s'appliqueraient quand même sous forme de décrets. Ce passage en force ne nous surprend pas au groupe communiste républicain et citoyen. Il n'est que la conséquence du parti pris à 100 % patronal, à 100 % MEDEF de l'exécutif Force est de constater que, sous couvert de modernisation, vous reprenez en fait une à une toutes les vieilles lunes du cahier des revendications patronales : primauté de l'accord d'entreprise, contournement des organisations syndicales, nouvelle réduction du champ du principe de faveur, facilitation et sécurisation des licenciements économiques, extension du travail de nuit et du dimanche, remise en cause du compte pénibilité, et j'en passe ! Ce sont autant de reculs des droits individuels et collectifs des salariés. salariés. Vous tentez de présenter cette énième réforme à une opinion publique mal informée comme une réponse aux bouleversements du travail, à la diversité des entreprises ou comme un levier pour dynamiser l'entrepreneuriat. Derrière l'imprécision du texte d'habilitation se cache, en réalité, une main de fer, celle qui est résolue à imposer la décentralisation des négociations collectives au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire là où le salarié est le plus en situation de faiblesse. Avec le principe de subsidiarité que vous sanctuarisez, vous inversez, en réalité, la hiérarchie des normes. Bien sûr, vous prétendez renforcer aussi le rôle des branches, mais hormis les domaines spécifiquement désignés par la loi ou les quelques possibilités de verrouillage, nombre de droits actuellement garantis par les conventions collectives de branche pourraient être remis en cause. Beaucoup s'en inquiètent, bien au-delà de notre sensibilité. Et en même temps, madame la ministre, vous recentralisez tous les pouvoirs entre vos mains en supprimant la commission d'experts prévue à l'article 1de la loi El Khomri, qui devait travailler à des propositions d'évolution du code du travail. Notre question préalable s'appuie sur ces données incontestables, mais plus encore sur le respect que nous portons à ces millions de Françaises et de Français précarisés qui cherchent un emploi ou qui voudraient simplement vivre décemment du leur. Le Président Le Président de la République a lui-même présenté ce texte comme un « préalable » à la modernisation de notre économie. Il n'y aurait donc pas de flexibilité dans la législation et la réglementation actuelles ? Permettez-moi d'en douter lorsque je vais sur la zone de Capécure, à Boulogne-sur-Mer, je m'aperçois que plus de 50 % des postes de production sont occupés en permanence par des intérimaires, qui ont sans doute des difficultés pour construire un projet de vie ou contracter un emprunt exemple, lorsque je téléphone dans mon département natal, la Manche, une ancienne voisine me dit tout ce qu'une société peut aujourd'hui imposer comme contraintes et obligations à un jeune pour gagner 230 euros à distribuer des annuaires téléphoniques ! Or le nombre des contrats « sauvages », ces CDD de moins d'un mois, est passé de 1,5 million en 2010 à 4 millions en 2016. doute les patrons ont-ils compris que ce serait encore mieux si le CDI lui-même était précaire ! Et c'est ce que vous nous proposez, d'une certaine manière Si je vous ai bien entendue, madame la ministre, il faut redonner confiance aux chefs d'entreprise pour recréer de l'emploi. Mais que faites-vous de toutes les études qui montrent qu'il n'y a pas de lien entre la protection de l'emploi et la montée ou la baisse du chômage ? L'ensemble des contre-réformes précédentes, dont les dernières remontent à l'année passée et qui n'ont d'ailleurs jamais été évaluées, n'a pas résolu le problème du chômage de masse en France. internationale du travail, la Banque mondiale et l'INSEE le démontrent, il n'y a pas de lien entre l'abaissement des droits et des garanties collectives et le règlement des problèmes de l'emploi et du chômage. C'est également vrai à l'échelle européenne, avec les mini-jobs à l'allemande, les contrats zéro heure à l'anglaise, le à l'italienne ou encore les reçus verts à la portugaise. pays ont-ils dégonflé artificiellement les statistiques du chômage, mais ils ont sûrement précarisé les travailleurs en plongeant nombre d'entre eux dans la misère, sans aucun effet réel sur l'emploi.

En réalité, c'est un projet de loi d'habilitation très politique, déconnecté des réalités, dangereux pour la performance de l'économie et notre équilibre social que le Président de la République vous demande d'autoriser, mes chers collègues, un texte qui va même au-delà des recommandations de la très libérale Commission européenne, laquelle saluait, dans les textes précédents- lois Macron, Rebsamen et El Khomri -, des « progrès substantiels

c'est construire un nouveau code du travail plus simple et plus protecteur, qui réponde aux défis du XXIsiècle, qui donne de nouveaux droits aux salariés et aux comités d'entreprise pour faire primer l'outil de travail sur la rapacité des fonds de pension prédateurs d'emplois ou les licenciements boursiers, un code du travail qui anticipe les mutations économiques, les évolutions technologiques, qui prenne aussi en compte les nouvelles aspirations des jeunes. La question des plateformes numériques, par exemple, n'est pas traitée dans ce texte. Pourtant, il est urgent de protéger les travailleurs concernés, et ce serait possible même en leur préservant une large indépendance, avec la définition

Ce remarquable travail, que vous ignorez malheureusement, madame la ministre, a été effectué par une vingtaine d'universitaires sous la direction d'Emmanuel Dockès, en concertation avec des syndicalistes de toutes les confédérations représentatives des salariés, sans exception. Mes chers collègues, parce que ce travail ne peut être ignoré, parce que le postulat sur lequel vous fondez ce projet de loi d'habilitation est manifestement erroné, parce que nous avons à coeur de défendre et le dynamisme de l'économie et la protection des salariés, je vous invite à voter la question préalable

opposer la question préalable. Nous pensons en effet que seuls le débat, l'expression d'opinions diverses, la confrontation des convictions, l'opposition des éventuelles argumentations font vivre, enrichissent et éclairent la démocratie.

souhaitent, et c'est leur droit, connaître les positions exprimées publiquement par leurs élus sur un projet de loi, fut-il d'habilitation, qui touche à une valeur fondamentale, le travail.

objectif d'accroître la compétitivité et l'attractivité de notre économie. Il vise aussi à simplifier, à rationaliser des dispositifs complexes issus d'une sédimentation de textes rendant le droit du travail parfois peu compréhensible, y compris d'ailleurs pour les spécialistes en la matière. Au final, de nombreux dispositifs n'offrent que des garanties formelles aux salariés, et non de réelles protections, tout en constituant une source de complexité juridique pour les employeurs.

Mme la ministre l'a expliqué la semaine dernière devant notre commission, la confiance des entrepreneurs repose sur une multitude de facteurs, au premier rang desquels figure le carnet de commandes. Vous le savez, mon cher collègue, l'économie, ce n'est pas que des statistiques, c'est aussi et surtout un état d'esprit. Nous devons donc créer un choc de confiance dans notre pays afin de redonner aux

préoccupation, c'est l'incertitude économique, leur capacité à décrocher des marchés, bien sûr, mais aussi les plans d'investissement et le soutien à l'investissement par la puissance publique. À cet égard, le plan d'investissement de 50 milliards d'euros

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande Le scrutin est ouvert.

les politiques des différents gouvernements qui se sont succédé durant cette période n'ont eu qu'un impact marginal sur la courbe du chômage. Il est évident que nous devons entreprendre des réformes et adapter notre droit du travail aux nécessités de notre époque. Pour reprendre vos propos, madame la ministre, lors de votre audition devant la commission des affaires sociales, il faut « libérer la dynamique de création d'emplois, tout en confortant les protections des salariés, réformées pour correspondre au monde d'aujourd'hui et de demain ». Les différents gouvernements, de droite comme de gauche, étaient bien sûr tous convaincus qu'ils détenaient la solution. Il faut avouer qu'ils ont rivalisé d'imagination pour mettre fin à ce fléau. Pourtant, force est de constater qu'ils n'ont pas réussi. Je pense tout particulièrement à mon île et à l'ensemble des territoires ultramarins, où le taux de chômage avoisine 25 %. Peut-être est-il temps d'observer chez nos voisins ce qui fonctionne. Vous avez également déclaré, madame la ministre, que vous recourriez aux ordonnances parce qu'elles articulent la démocratie politique- grâce au débat au Parlement sur les projets de loi d'habilitation puis de ratification ratification -, et la démocratie sociale, ce qui est bien le moins pour un projet de loi dont l'objet est de renforcer la démocratie sociale. Je me félicite bien évidemment que vous ayez respecté l'article L. 1 du code du travail, cher au président Larcher, concernant les modalités de concertation des partenaires sociaux sur toute réforme, contrairement à votre prédécesseur ! Je ne peux cependant pas en dire de même concernant votre choix de recourir aux ordonnances, sur un texte de cette importance, d'abord par principe. Les ordonnances constituent une forme de « législation déléguée qui affaiblit le rôle du Parlement, au même titre qu'une interprétation trop restrictive du droit d'amendement ou le recours systématique à la procédure accélérée. Ce faisant, elles renforcent les postures manichéennes au lieu d'exploiter la force de proposition des parlementaires. Ce n'est pas notre vision du travail législatif. Chacun devrait se rappeler étaient à l'origine une procédure exceptionnelle destinée à faire face à une situation urgente et pour un délai limité seulement, comme le soulignait l'avant-projet constitutionnel en date du 29 juillet 1958. En 2005, dans un retentissant article, dont chacun se souvient, intitulé, le professeur Delvolvé avait à juste titre critiqué un « dérèglement juridique et politique » s'étant progressivement étendu à des pans entiers du droit, en premier lieu au droit de l'outre-mer. Année après année, nous constatons que ces mauvaises habitudes estivales ont la vie dure dure ! Nous voyons ainsi d'un mauvais oeil le fait que le Gouvernement y ait recours dès ses premières semaines au pouvoir, sans que l'urgence soit véritablement caractérisée. Dans le cas particulier de dispositions sur les conditions de travail, nous pensons que cela conduit à remplacer la démocratie parlementaire par la démocratie sociale, plutôt que de les articuler entre elles. Certes, ce projet de loi d'habilitation est conforme à l'engagement pris pendant la campagne du Président de la République qui souhaitait légiférer par ordonnances « pour des raisons d'efficacité et de rapidité ». Pour autant, et le rapporteur l'a très justement rappelé, le champ de ce projet de loi d'habilitation est extrêmement vaste et certains aspects auraient pu être traités ultérieurement, et non dans des délais particulièrement courts alors même que la concertation avec les partenaires sociaux doit se poursuivre au moins jusqu'à la fin du mois de septembre. l'ensemble du moins la majorité des sénateurs, sont réticents au fait de signer un chèque en blanc au pouvoir exécutif, quel qu'il soit, surtout d'une réforme d'une telle ampleur. Pour obtenir le feu vert du Parlement, le Gouvernement se doit d'être plus précis. Aussi, j'espère, madame la ministre, que vous comprendrez la nécessité d'apporter des précisions au cours de nos débats.

dont l'application risque d'entraîner, il faut bien le reconnaître, quelques difficultés, mais qui représente un progrès social majeur pour les salariés exposés à des travaux pénibles. Pour autant, nous déplorons la démarche

Ce n'est pas acceptable. Madame la ministre, nous devons absolument nous fixer pour un objectif de permettre aux salariés exposés à des travaux pénibles de partir en retraite en bonne ou assez bonne santé Par ailleurs, comme l'a rappelé Gilbert Barbier en commission, « la lettre du Premier ministre aux partenaires sociaux atteste de ce manque de prise en compte de la prévention des risques. Se contenter d'une visite médicale en fin de carrière

favorables au texte adopté par l'Assemblée nationale, la majorité de notre groupe ne pourra apporter son entier soutien à la version présentée par notre commission des affaires sociales, qui marque, il nous semble, un recul pour les droits des salariés. Je pense en premier lieu aux modifications apportées à l'article 1, et principalement à la représentation des salariés dans les petites entreprises, notamment celles de moins de cinquante salariés. Vous l'avez rappelé devant la commission, « sous ce seuil, où travaillent 55 % des salariés, seulement 4 % des entreprises disposent de délégués syndicaux ou de représentants du personnel mandatés par une organisation syndicale, ce qui revient à dire que le dialogue social ne peut aboutir à des accords d'entreprise, alors qu'on a particulièrement besoin de souplesse dans ces entreprises Je regrette également la version adoptée en commission, qui prévoit notamment de contourner les organisations syndicales en permettant aux employeurs dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de délégué syndical de conclure des accords collectifs directement avec les représentants du personnel et, en leur absence, directement avec le personnel. Le texte dont nous allons débattre est un projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

à ces salariés d'avoir accès au dialogue social. Je pense qu'il faut vous laisser le temps de trouver un dispositif qui réponde aux spécificités des petites entreprises. Concernant l'article 3, relatif à la sécurisation des relations de travail, la commission des affaires sociales a adopté plusieurs modifications qui ne nous semblent pas aller dans le bon sens, telles l'instauration du droit à l'erreur au bénéfice de l'employeur pour lui permettre de rectifier des irrégularités en matière de motivation dans la lettre de licenciement ou la réduction à six mois du délai de recours recours sur la régularité ou la validité d'un licenciement pour motif économique. Madame la ministre, vous l'aurez compris, les sénateurs du RDSE seront particulièrement attentifs aux débats

le compte personnel d'activité, la commission paritaire régionale interprofessionnelle, les accords de prévention et de développement de l'emploi, et tout un ensemble d'autres inventions administratives. Le code du travail n'a cessé d'enfler ... Cela me désespère. Les entrepreneurs, eux, sont exaspérés. Parfois, ils sont contraints de trouver des accords avec leurs salariés en dehors de la loi ... jusqu'au jour où ces derniers changent d'avis.

D'autres entrepreneurs, comme moi, veulent une vie simple et sereine. Ils préfèrent s'affranchir de toutes les règles franco-françaises et d'un coût du travail qu'ils jugent exorbitant. Ils font le choix d'entreprendre ailleurs. Il y a deux ans, je proposais, un amendement au projet de loi dit Macron, de modifier l'article L. 1 du code du travail pour inverser la hiérarchie des normes. À l'époque, alors que l'on me demandait de retirer mon amendement en séance, j'avais déclaré que je voulais qu'il soit mis aux voix « pour l'histoire ». Je refusais un droit du travail qui allait à contre-courant de ce qui est la norme des pays performants.

Un an plus tard, soit l'année dernière, le rapport de M. Combrexelle a fait admettre la nécessité de cette inversion. Dans tous les pays qui ont une compétitivité forte, le code du travail est réduit et la place de la négociation collective est prépondérante. La loi El Khomri a engagé le retournement que j'avais préconisé. Madame la ministre, je me réjouis des perspectives tracées dans votre projet de loi, qui me permettent d'espérer que vous allez poursuivre dans cette voie ; j'y reviendrai. Quel dommage Quel dommage que, à l'époque, le ministre Emmanuel Macron n'ait pas fait adopter mon amendement : nous aurions gagné beaucoup de temps ... Faut-il aujourd'hui une nouvelle réforme du droit du travail ? Oui, car le chômage est toujours aussi important et la relance économique encore timide. Il est urgent de donner du souffle au monde du travail et de libérer les énergies. Notre droit du travail est devenu obsolète : il faut l'adapter aux nouveaux enjeux d'une économie mondialisée et dématérialisée, en donnant aux salariés les moyens de faire évoluer leur carrière tout en protégeant les plus fragiles.

Voilà maintenant un an, à la même époque, nous venions de terminer deux semaines de discussion du projet de loi El Khomri : plus de 1 000 amendements déposés, des jours et des nuits en séance à nous opposer ; au même moment, dans la rue, les manifestations et violences épuisaient nos concitoyens. La majorité sénatoriale avait proposé une version plus ambitieuse d'un texte qui, dès le départ, n'avait pas été pensé et présenté pour réussir. Si le gouvernement d'alors avait voulu l'échec de sa réforme, il ne s'y serait pas pris autrement Le recours aux ordonnances se justifie : au Parlement de donner un périmètre, au Gouvernement de concrétiser cette réforme. La discussion du projet de loi de ratification sera l'occasion de vérifier que le périmètre a été respecté. Il faut aller vite afin que les effets apparaissent. En parallèle, le Gouvernement paraît vouloir corriger les erreurs de son prédécesseur, lequel n'avait pris le temps ni la peine de présenter sa réforme et de négocier avec les partenaires sociaux. Beaucoup ici, sur les travées de la gauche, avaient alors justifié cette façon de procéder. Rien de tout cela aujourd'hui. Les nombreux rendez-vous pris entre vous, madame la ministre, et les partenaires sociaux témoignent d'une volonté d'associer ces derniers Vous aurez ici, au Sénat, l'occasion de débattre, de coconstruire pour enrichir le texte voté à l'Assemblée nationale, où les discussions ont semblé bien timides aux observateurs. Nous soutenons le principe du recours aux ordonnances en matière de droit du travail, car nous l'envisageons comme la première étape d'une série de réformes nécessaires et urgentes anticipées par le Gouvernement, portant sur la formation professionnelle, l'assurance chômage, les retraites. Les ordonnances sur le droit du travail ont pour objectif de flexibiliser le marché du travail en donnant plus de place à la négociation d'entreprise. Le volet relatif à la protection et à la sécurité des salariés devra principalement se retrouver dans les réformes à venir : celles de la formation professionnelle pour adapter ses compétences et de l'assurance chômage pour les phases de transition. Cette vision d'ensemble conforte notre soutien. Pourquoi est-il incontournable de rénover notre droit du travail ? Il n'a échappé à personne- quoique, pour certains, j'en doute ! -que l'économie a changé depuis le tournant du siècle. Nous sommes au début d'une ère numérique, à l'aube de la troisième révolution industrielle, dans laquelle coexisteront et se développeront les,, et autres. Ces nouvelles technologies transforment les métiers. Il faut cultiver des compétences transversales au coeur de métiers hybrides. Les collaborateurs devront être autonomes grâce à un travail en parallèle et interactif, s'affranchissant du temps et de l'espace. Cette révolution numérique se fait au coeur d'une économie mondialisée. Les échanges sont globaux, de plus en plus rapides, les frontières disparaissent. Puisque je suis un sénateur-entrepreneur, je partagerai mon expérience personnelle. Toutes les personnes qui contribuent à mon entreprise établie au Royaume-Uni sont des travailleurs indépendants : elles m'offrent leurs compétences depuis leur domicile, elles sont localisées aux quatre coins de la planète, elles s'organisent comme bon leur semble, travaillent au moment où elles le souhaitent. Plus jamais on ne me demande si elles peuvent partir en vacances ou quand. Seul le résultat compte. Vouloir être libre, c'est vouloir les autres libres. Nous devons faire émerger un nouveau droit du travail qui encourage le dialogue social et économique, un droit qui prenne en compte les nouvelles formes de télétravail, ces exigences d'autonomie, ces parcours individualisés. Si nous voulons attirer les entrepreneurs qui vont quitter le Royaume-Uni à la faveur du Brexit, il va falloir révolutionner notre système Il va falloir replacer le droit du travail au coeur des besoins des entreprises et de leurs salariés. Il va falloir libérer les énergies ! Ce sont ces objectifs qui doivent guider votre réforme, madame la ministre. Vous devez aller vite, mais vous devez surtout aller loin. Les ordonnances vont vous permettre d'aller vite,

Jusqu'où irez-vous pour placer le dialogue social au plus près des salariés et de leur entreprise ? L'article 1 de votre projet consacre une nouvelle fois l'inversion de la hiérarchie des normes que j'ai évoquée. Irez-vous jusqu'au bout ou allez-vous prévoir tellement d'exceptions que ce sera une nouvelle réforme pour rien ? Vous devez replacer à l'échelon de l'entreprise, du groupe ou de la branche l'ensemble des règles applicables en matière de droit du travail et de formation professionnelle. La France est, avec la Belgique, l'Espagne et la Grèce, l'un des derniers pays à accorder une place prépondérante à l'État dans le dialogue social. Vous devez faire confiance aux partenaires sociaux en choisissant de les responsabiliser. De ce point de vue, vos propos m'ont réjoui. Quant à la loi, son rôle s'inscrira dans le cadre strict de l'article 34 de la Constitution : le législateur continuera de fixer les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la protection sociale. Jusqu'où irez-vous pour améliorer le dialogue social dans les entreprises ? La généralisation proposée d'une instance unique de représentation des salariés sera une excellente avancée. Mais oserez-vous faire encore plus confiance aux salariés, en leur permettant de négocier directement dans certaines entreprises ? La France est l'un des derniers pays de l'Union européenne pour le taux de syndicalisation. Maintenir à ce point le monopole des syndicats dans le dialogue social

Le marché du travail est si tendu dans ce pays que les employeurs font le maximum pour conserver leurs collaborateurs. Il faut également et impérativement s'attacher à supprimer les effets de seuils, qui posent un vrai problème aux entreprises de notre pays. Ces seuils ne créent pas uniquement des difficultés en matière de mise en place des délégués du personnel avec les obligations qui en découlent, ils augmentent aussi fortement les coûts pour les TPE. Il faut au minimum relever les seuils fixés à 10 et à 50 salariés. J'avais proposé de nous en tenir aux seuils européens de 50 et 250 salariés. Ces mesures sont compatibles avec l'instauration d'un dialogue social au plus près des salariés, directement, sans intermédiaire,

Chez nos voisins d'Europe du Nord, la simplification est un objectif politique transpartisan. Elle répond à une méthodologie rigoureuse, qui repose sur des objectifs et sur le suivi d'indicateurs. En Allemagne, aux Pays-Bas et en Suède, un organe indépendant contrôle la qualité des études d'impact. Pourquoi ne pas s'inspirer de leur exemple ? Les entreprises étouffent sous le poids des procédures administratives : plus personne n'y comprend rien. C'est la conséquence de l'inflation de normes, qui noie les entreprises

Pourtant, notre industrie du raffinage connaît plus d'accidents que la moyenne européenne : les raffineries françaises concentrent 26 % des accidents en Europe, alors qu'elles ne représentent que 10 % des sites. Comment ne pas évoquer ici la médecine du travail ? À l'heure actuelle, environ 80 % des salariés travaillent dans le secteur tertiaire. Leur médecin traitant, qui les connaît depuis des années, ne serait-il pas compétent pour juger s'ils peuvent travailler assis derrière leur bureau ? Pourquoi vouloir maintenir une médecine administrative ? Le médecin du travail serait-il un spécialiste de toutes les maladies que l'on peut attraper en travaillant ? Nous devons nous demander si ce système est encore adapté à la grande majorité des salariés et s'il les protège réellement.

Jusqu'où irez-vous pour flexibiliser le marché du travail ? Vous proposez de fixer un barème des dommages et intérêts, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Comment justifier, en effet, qu'il y ait, pour un même préjudice, des différences aussi importantes entre deux conseils de prud'hommes ? Comment justifier que le licenciement d'un salarié puisse, à lui seul, mettre en péril une entreprise, tant les indemnités demandées sont parfois colossales ? Pense-t-on aux autres salariés ? J'avais déposé des amendements visant à plafonner les licenciements économiques, que le juge contrôle le périmètre des difficultés, mais en aucun cas l'opportunité de licencier ! Une entreprise est libre de décider de créer un département et de recruter une équipe pour lancer un nouveau produit ; elle doit être tout aussi libre de le fermer et de licencier en cas d'échec commercial. Le juge ne doit pas avoir la faculté d'apprécier cette décision et, éventuellement, de la remettre en question. Mais bien sûr ... Nous sommes tellement bavards en élaborant le code du travail, nous avons tellement le souci de tout prévoir que nous créons nous-mêmes les futures chausse-trappes en omettant des situations. La liquidation judiciaire n'étant pas expressément visée par un article de la loi El Khomri, cela permet aux salariés de remettre en cause le motif économique de leur licenciement, quand bien même ce motif est lié à une décision du juge-commissaire ou du tribunal de commerce. Je ne sais pas si chacun a bien conscience du point où nous en sommes : une liquidation judiciaire n'interdit pas à un salarié de contester son licenciement économique. C'est le pays d'Ubu Je ne parle même pas de la longueur des procédures : pendant plusieurs mois, les entreprises sont contraintes de payer un salarié qui ne travaille déjà plus ! Il faut enfin aller beaucoup plus loin sur les modalités de recours aux CDD, en en allongeant la durée maximale, instaurer un CDI à droits progressifs et prévoir que celui-ci puisse prédéfinir les motifs et conditions de sa rupture. Je suis convaincu qu'une réforme profonde du droit du travail, allant dans le sens d'une plus grande rapidité en matière d'embauche et de fin de contrat, aurait une incidence directe sur le nombre de défaillances d'entreprises dans notre pays, à conjoncture économique égale. Des administrateurs judiciaires témoignent avoir vu nombre d'entreprises mourir de ne pouvoir mettre en place un plan social rapidement confrontées à des procédures prud'homales hors de proportions avec leurs capacités, s'agissant en particulier des TPE. On peut même envisager qu'une telle réforme ait un impact positif sur la conjoncture elle-même Jusqu'où irez-vous pour simplifier l'organisation du travail ? Vous proposez de réfléchir aux nouvelles formes de travail, en favorisant l'accès au télétravail et au travail à distance. C'est un objectif essentiel : vous devez assouplir au maximum les règles permettant aux salariés d'y recourir et ne surtout pas entrer dans un système de contrôle administratif impossible à mettre en oeuvre. Jusqu'où irez-vous, madame la ministre ? À la fin des années quatre-vingt, le PDG de la société Sun Microsystems a demandé à ses ingénieurs de faire rentrer l'informatique des ordinateurs les plus puissants, qui occupait une armoire, dans un volume équivalent à celui d'une boîte à pizza. Il a révolutionné son industrie. Nous avons besoin de révolutionner notre code du travail, de le rendre simple, lisible et compréhensible par tous.

En recourant à des ordonnances, vous prenez la responsabilité entière des décisions à venir et de leurs conséquences pour les entreprises et notre économie. Parce que, foi de Jupiter, Rome ne s'est pas faite en un jour,

principe à l'utilisation des ordonnances, pratique dérogatoire qui, parce qu'elle est dérogatoire, demande à être parfaitement justifiée.

la loi El Khomri visait à améliorer la capacité d'adaptation des entreprises aux cycles économiques et les conditions de travail. Situation surréaliste, pendant que nous débattions en commission, les auditions des partenaires sociaux se poursuivaient, apportant leur lot de propositions auxquelles nous n'avions pas accès. procédure inédite et contraire au principe de la démocratie parlementaire ... Très bien ! Le 49-3, si décrié, est-il si éloigné de cette procédure ? Ainsi, ratifiées ou non, les ordonnances, à l'élaboration desquelles nous n'aurons pas participé, seront applicables et, n'en doutons pas, seront appliquées en qualité de loi ou, à défaut, de texte réglementaire. Curieuse procédure ! Ni l'urgence ni une nécessité absolue ne sauraient justifier ici la dépossession du Parlement de ses prérogatives. Doit-on en déduire que le dialogue brandi comme méthode de gouvernement n'est qu'une illusion ? Pour l'heure, je me garderai bien de conclure. Venons-en au contenu. Convenons qu'il est difficile, devant un projet aux orientations tellement vagues- si belles et si généreuses soient-elles dans leur libellé -, de se faire une opinion précise. Il faut aller chercher dans les déclarations auprès des organisations syndicales et professionnelles des bribes d'information qui, bien qu'indirectes, nous renseignent mieux sur les intentions réelles du Gouvernement. C'est donc souvent par ce qu'on devine de subliminal ou d'inscrit en filigrane que nous avons pu cerner un peu mieux le devenir de ces ordonnances. La tentation aurait pu être grande de rejeter d'emblée la proposition pour « cause de vide ». Nous n'y avons pas cédé et avons souhaité apporter notre vision- déjà exprimée antérieurement -d'une modernisation fructueuse et dynamique du code du travail. Le Gouvernement était guidé, était-il annoncé, par deux ambitions. La première était de donner à nos entreprises de la compétitivité. Les indicateurs économiques affichant enfin une belle couleur verte, les nouvelles dispositions donneraient un coup de pouce supplémentaire à la croissance retrouvée. La seconde ambition se dégageait des grandes déclarations : assurer aux salariés une plus grande sécurité dans un monde qui se transforme, s'engage dans le numérique, bouleverse la structure de l'emploi, exige le suivi de formations tout au long de la vie, droit qui doit être renforcé pour ceux dont la formation initiale est la plus légère, ce que la loi El Khomri avait largement pris en compte. Mais faute d'évaluation Or, si la première ambition de renforcer la compétitivité est bien servie, il apparaît clairement que la sécurisation des parcours professionnels, la reconnaissance syndicale ont été largement sacrifiées sur l'autel du libéralisme. Les amendements d'une droite fondue dans une majorité de circonstance ont encore aggravé le déséquilibre. Je me contenterai, pour l'heure, de prendre quelques exemples particulièrement édifiants des intentions du Gouvernement et de la commission, qui ne laissent pas de nous inquiéter. six mois des délais de recours pour les salariés contre des décisions les concernant, certains d'entre eux, peu familiers des procédures juridiques, éprouveront des difficultés à agir dans les temps. La présomption

type de licenciement, mais le risque est grand de faire du licenciement une banale formalité administrative. Licencier est un acte dramatique, qui peut détruire toute la vie du travailleur et celle de sa famille. C'est un acte grave auquel nombre de chefs d'entreprise ne se résolvent que douloureusement et qui nécessite un peu plus d'humanité que le fait de renseigner un simple imprimé. du licenciement, qui viendrait remplacer les formes actuelles, se traduira par des indemnisations inférieures à celles qui sont attachées à un licenciement économique. La fixation d'un plafond pour la compensation du préjudice subi du fait d'un licenciement apparaît particulièrement inacceptable et constitue une grave entorse à un principe fondamental de notre droit qui exige que tout jugement soit individualisé.

Que dire des atteintes aux conditions de travail que constituent l'extension et la banalisation possible par accord d'entreprise du travail de nuit, lequel, aux termes de notre législation, doit toujours être considéré comme exceptionnel On ira même jusqu'à utiliser la sémantique avec une délicieuse subtilité pour qualifier de CDI « de chantier » ou « de mission » des contrats dont la durée est limitée

l'obtention d'un prêt ou la location d'un logement. Ainsi sont satisfaites les demandes patronales largement puisées dans le rapport « Propositions pour reconstruire la négociation sociale » de l'Institut Montaigne de Claude Bébéar et Henri de Castries. Enfin, sont inacceptables les nouvelles dispositions sur la pénibilité. Six domaines ont été retenus sur les dix qu'avait définis le gouvernement Ayrault. Certes, les quatre autres sont difficiles à apprécier. Pour autant, abandonner toute démarche préventive pour se contenter de mesurer les dégâts au moment du départ à la retraite, c'est refuser de réduire cette injustice intolérable que constitue la moindre longévité en moins bonne santé d'un certain nombre de nos concitoyens confrontés à des risques lourds. Même si résoudre le problème posé n'est pas facile, c'est un devoir ardent et urgent d'en trouver la solution et de la mettre en oeuvre. J'ose espérer que les ordonnances sauront apporter des réponses fondées sur la prévention des maladies et handicaps invalidants. Je m'en tiendrai là sur ce sujet. La discussion nous permettra d'aller plus avant et d'alerter sur les conséquences toxiques des mesures qui se dessinent au travers de ce projet de loi d'habilitation, lourdement aggravées par les propositions de la commission des affaires sociales.

entre le chef d'entreprise et le délégué du personnel, voire par interrogation directe du personnel. C'est en parfaite contradiction avec la volonté de développer l'audience des organisations syndicales ! Tout à fait ! Dans la situation de subordination qui est une négociation ne peut être menée de façon équilibrée quand le signataire désigné peut toujours craindre des représailles. Même s'agissant des entreprises où le dialogue est aisé, serein, constructif, penser que la négociation puisse être menée sans crainte et sans autocensure relève de la fiction. Angélisme ou machiavélisme, peu importe : la régression sociale risque d'être au bout du chemin. La fusion de toutes les instances représentatives du personnel

Cependant, la commission veut réduire le nombre de mandats consécutifs, ce qui va à l'encontre de l'acquisition des compétences nécessaires. Très bien ! Il faut laisser leur spécificité et la personnalité morale aux CHSCT, qui traitent de sujets essentiels- la santé, les conditions de travail -dans un monde qui va inévitablement voir se multiplier les risques sanitaires. L'exercice de ces responsabilités nécessite une grande indépendance par rapport aux considérations économiques : pensons au scandale de l'amiante. Le CHSCT, ou son ersatz, doit conserver la personnalité morale qui confère le droit d'ester. Ainsi, au-delà des intentions déclarées, certaines propositions, issues notamment des votes de la commission, sont attentatoires à la qualité du débat dans l'entreprise, débat d'autant plus nécessaire que s'instaure avec force la primauté

la CSG pour les retraités, renforcement des inégalités ... Ici également, on constate un grand écart entre les ambitions affichées et la réalité qui s'annonce. Madame la ministre, les partenaires sociaux ont été favorablement impressionnés par la qualité d'écoute que vous avez montrée. Soyez-en félicitée : c'est une attitude louable pour un élu, pour un ministre. Mais il ne faudrait pas vous en tenir là. Plaisir d'amour, » dit la chanson, « ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie. » Après le plaisir de la rencontre, souhaitons que les ordonnances à venir ne soient pas porteuses de grandes déceptions. C'est, hélas, ce qui s'annonce. Personne ne souhaite l'échec du Gouvernement, pour des raisons que tout le monde comprendra.

Ne croyez-vous donc pas que, pour lutter contre le fléau du chômage, plutôt que de bricoler- certains diront détricoter -le code du travail, il faudrait changer de modèle de développement, changer de politique économique ? Cela fait quarante ans que vous essayez de corriger les dérives de ce modèle sans y parvenir. Je suis persuadé que, tout comme le modèle communiste s'est effondré,

Avec ce modèle, votre modèle, pendant que les salariés grecs, sur injonction de Berlin, étaient payés en tickets restaurant, l'économie allemande gagnait 100 milliards d'euros ! Les puissances d'argent ont pris le pouvoir économique et l'économie est devenue une fin en soin au lieu d'être un moyen au service de l'humain, au service de la vie en société. Cela se traduit notamment dans le dialogue social, sujet de ce texte : syndicats de salariés comme syndicats patronaux ne recherchent plus un bien commun qui les dépasserait ; non, ils cherchent avant tout à exister C'est ce qui fait qu'ils sont si peu considérés par les Français, qu'ils sont si peu représentatifs ! Alors, avant de réformer le dialogue social, il eût mieux valu commencer par réformer les « dialogueurs », si vous me permettez ce néologisme. Ce n'est pas le chèque syndical déguisé que l'article 2 vous permettrait d'instaurer qui conduira les syndicats à se préoccuper du bien commun des salariés plutôt que de leur seul intérêt.

au service d'une société plus juste. Il ne fait, en réalité, qu'accompagner un modèle économique qui, depuis quarante ans, montre d'année en année ses limites ! Comment peut-on, lorsqu'on a la défense du bien commun chevillée au corps, comme c'est, j'en suis persuadé,

ces milliardaires ne font pas des affaires qu'en France, mais la captation de la totalité de la croissance créée par la France en une année par seulement trente-neuf personnes ne vous émeut manifestement pas beaucoup ! En réalité, ce texte symbolise très bien l'obstination dans un modèle voué à un triple échec. Échec social, d'abord, car les salariés vont devenir plus que jamais, pour les entreprises,

entre salariés et employeurs, cassant les relations existant aujourd'hui entre salariés et employeurs, certes imparfaites et fondées inévitablement sur un aspect pécuniaire, mais tout autant sur une adhésion à un projet collectif, sur la confiance, sur la solidarité et, bien sûr, dans la mesure du possible, sur la durée. Pourquoi encourager la marchandisation de toutes les relations humaines ? Échec économique, ensuite, car ce texte n'aidera en rien les PME et les TPE qui forment la majeure partie du tissu entrepreneurial de notre pays

soient au service de l'homme et du bien commun, il me semble nécessaire qu'elles conservent une taille humaine. D'ailleurs, le dialogue social, même s'il y est moins codifié, est souvent bien meilleur dans les petites entreprises que dans les grands groupes. En effet, à cette échelle, on vit ensemble, on se serre les coudes, on gagne des marchés ensemble, on monte des projets ensemble, on innove ensemble et on fait face aux difficultés ensemble Une vraie simplification administrative et une vraie baisse des charges pour les PME, les TPE et les artisans, voilà l'urgence ! Votre collègue M. Bruno Le Maire nous a parlé la semaine dernière d'un texte en préparation ; espérons qu'il soit axé sur ces deux volets ! Échec écologique,

nous ne voterons pas ce texte, parce qu'il consacre l'idée d'une société nomade, d'une société de déracinés où les relations humaines reposent d'abord sur l'argent, les salariés devenant des mercenaires interchangeables.

nous a dit le Président de la République lors du Congrès qui nous a réunis à Versailles, le 3 juillet dernier. Puisque nous sommes en période révolutionnaire, il ne faut pas s'étonner que nous utilisions des moyens inédits et que nous empruntions des chemins nouveaux. aux ordonnances pour agir vite : notre pays en a vraiment besoin.

sociaux. Il faut se réjouir que, pour une fois, la démocratie sociale et la démocratie parlementaire cheminent côte à côte.

Prenons donc ces ordonnances pour ce qu'elles sont, le volet initial de réformes radicales qui vont se succéder durant ce quinquennat : celles de l'assurance chômage, de la formation professionnelle

pour accompagner la mutation des métiers et des technologies. Il nous faut élever globalement le niveau de compétences et mobiliser toutes les parties prenantes de l'entreprise afin de préparer et d'accompagner les choix stratégiques

Dans le champ conventionnel, le choix est clairement fait de mener ce dialogue au plus près des acteurs, c'est-à-dire dans l'entreprise, en élargissant son périmètre tout en confortant le rôle de régulation

notamment des jeunes, lesquels payent aujourd'hui au prix fort, celui de la précarité, leur entrée dans la vie professionnelle. Le Gouvernement a donc eu raison d'avoir placé en haut de l'agenda de la session extraordinaire

Malheureusement, le texte de la commission ne s'est délivré ni des unes ni des autres. La majorité sénatoriale y a introduit, comme l'a souligné l'un de nos collègues

laissez-les vivre, quand même ! À l'article 3, qui traite des licenciements économiques, vous donnez mandat impératif au Gouvernement en vue de la ratification. Vous imposez

C'est pour laisser le maximum de chances de parvenir à des compromis positifs que le champ des ordonnances, tel que défini par le Gouvernement et modifié à la marge par l'Assemblée nationale, est volontairement large. Cela permet de balayer tous les sujets qui concernent le travail

en commission, habilite le Gouvernement à « déterminer les conditions dans lesquelles les représentants du personnel peuvent être mieux associés aux décisions de l'employeur

que le dialogue social aura une assise encore plus solide si les choix stratégiques des entreprises sont mieux partagés. Je rappellerai, à ce sujet, que la loi Rebsamen avait abaissé les seuils des effectifs

Nous ne pouvons rester parmi les rares pays affichant un tel niveau de chômage. Nous devons tirer les conséquences de la mondialisation, mesurer avec lucidité les mutations technologiques. Il faut s'en saisir, ne pas les subir. Il y a, dans notre beau pays, une aspiration à la liberté dans l'économie, dans les parcours de vie, et une attente de protection nouvelle face à ces changements. Qui peut contester ici un tel objectif ? La question est la suivante : comment comptez-vous, madame la ministre, réussir ce beau projet ? Malheureusement, votre réponse va à l'encontre de l'objectif affiché, puisque vous voulez réduire les droits des salariés, faciliter le recours aux contrats précaires et aux licenciements et supprimer, autant que faire se peut, les obligations des grandes entreprises. Vous dites vouloir faire de la politique autrement- autrement- M. Macron a même été élu sur cette promesse -, mais, dans les faits, vous poursuivez la politique libérale qui a été menée dans notre pays, depuis trente ans, par vos prédécesseurs et dont nous ne connaissons malheureusement que trop bien les conséquences. « Il faut que tout change

il y a, en réalité, une volonté de justifier votre projet idéologique de casser notre pacte social. Au nom de la modernité, tous les acquis sociaux devraient disparaître. Ainsi, être moderne, c'est autoriser les employeurs à licencier contre un chèque équivalent à vingt mois de salaire Être moderne, c'est mettre en oeuvre un CDI précaire, limiter le pouvoir des juges pour augmenter celui des employeurs. Être moderne, c'est supprimer les représentants syndicaux, qui contestent les plans de licenciement. Pour la majorité présidentielle, les archaïques sont donc celles et ceux qui se préoccupent de la prise en compte réelle et effective de la santé des salariés, notamment en défendant la prévention au travers du maintien des CHSCT, dont le rôle de contrôle spécialisé des conditions de travail, de sécurité et de santé au sein de l'entreprise est primordial. Les archaïques sont celles et ceux qui pensent que la représentation des salariés dans l'entreprise est nécessaire pour défendre leurs droits et que les syndicats sont un rempart démocratique pour négocier à égalité avec les employeurs. Alors, je suis fière, mes chers collègues, comme chacun des membres de mon groupe, d'être archaïque ! Tout à fait ! Derrière le mot d'ordre « modernité », quel est le modèle que vous souhaitez mettre en place ? Est-ce celui de la « flexisécurité » à la danoise, qui allierait une plus grande facilité de licenciement et une bonne indemnisation des demandeurs d'emploi ? Depuis les années quatre-vingt-dix, il a pourtant été démontré que la flexibilité des droits prend largement le pas sur la sécurité des salariés. Nous avons vu, lors de la crise de 2008, que ce modèle a moins bien résisté que le nôtre ; on a observé au Danemark une forte hausse du taux de pauvreté, notamment chez les jeunes. En réalité, en France, la flexisécurité existe depuis longtemps. Comme le dénonce l'économiste Anne Eydoux, « dans les années 1980, lors de la réforme du temps partiel, le Gouvernement avait assuré que cette mesure allait enrichir la croissance, en amenant les femmes à l'emploi. Sauf que le taux d'emploi des femmes a à peine augmenté

Madame la ministre, mes chers collègues, je suis au regret de vous dire qu'asservir les salariés en augmentant à votre guise leur temps de travail, en dégradant leurs conditions de travail ou encore en diminuant librement leur salaire, n'a rien d'un modèle et n'est en rien moderne. Vous mettez en avant, comme contrepartie de la flexibilité, une sécurité renforcée pour les travailleuses et les travailleurs. La sécurité des salariés, à vos yeux, consiste donc à remplacer le compte de prévention de la pénibilité par un compte de réparation. La sécurité, c'est enfin, selon vous, la barémisation des dommages et intérêts, qui permettra aux employeurs de connaître à l'avance le prix d'un licenciement abusif, et donc de l'organiser. Affaiblir le droit du travail pour promouvoir la négociation s'inspire aussi du modèle nordique, alors même que la construction du dialogue social est très différente dans notre pays. Contrairement au système de cogestion danois, la France a en effet inscrit les obligations de négocier dans le droit. Le Gouvernement veut privilégier les accords d'entreprise au détriment des accords de branche. Mais aujourd'hui, dans les TPE, où il n'y a pas de représentants du personnel, ce sont les accords de branche qui servent de protection. Pourquoi l'ignorer ? De bien mauvaise foi sont ceux qui nient aujourd'hui le lien de subordination existant entre un employeur et ses salariés. Vous pouvez le supprimer dans tous les textes que vous voudrez, il n'en cessera pas moins d'exister.

en autorisant notamment les entreprises de moins de 50 salariés à s'affranchir tout bonnement de l'obligation de négocier avec les représentants du personnel. Gardons à l'esprit, mes chers collègues, que 95 % des entreprises ont moins de 50 salariés. Cela voudrait donc dire que, à l'avenir, 95 % des salariés ne bénéficieront plus d'aucune protection collective. Non seulement cette liquidation en règle du code du travail ne réglera pas le problème du chômage, mais elle aggravera les conditions de travail dans les entreprises. Elle occasionnera, baisses de productivité, au rebours de ce que l'on est en droit d'exiger au XXI siècle. Libérer le travail, c'est au contraire, pour nous, lui redonner du sens, c'est soutenir la créativité des salariés, c'est mettre l'humain au coeur de l'entreprise en donnant des pouvoirs nouveaux aux salariés sur tout ce qui a trait à leurs conditions de travail mais aussi, plus largement, à la gestion même de l'entreprise. Libérer le travail, c'est assurer la sécurisation des parcours professionnels à travers l'emploi et la formation, comme nous le préconisons au moyen d'une proposition de loi. Mes chers collègues, ne vous y trompez pas : le Gouvernement est parfaitement conscient d'opérer un hold-up législatif, sinon il n'agirait pas à ce point dans l'urgence. S'il y a urgence, c'est que le Gouvernement est conscient qu'un tel texte ne serait pas passé si facilement dans le cadre d'un processus législatif normal. Personne n'est dupe. Je me permettrai de pointer qu'il est tout de même assez cocasse de prétendre renforcer le dialogue social en passant par des ordonnances qui musèlent le Parlement. Très bien ! Le Gouvernement cherche délibérément à profiter des congés d'été des Françaises et des Français- congés payés acquis de haute lutte lors du Front populaire, faut-il le rappeler -pour empêcher toute mobilisation syndicale, toute manifestation d'envergure. La période estivale est évidemment propice à de telles manoeuvres. Il faut d'ailleurs croire qu'avec ce nouveau gouvernement, avec l'Assemblée nationale fraîchement élue et majoritairement aux couleurs du Président de la République, dont tout le monde feint d'avoir oublié qu'il a été un ministre zélé de François Hollande, la flexibilité ne doit s'appliquer qu'aux seuls salariés, en aucun cas au texte gouvernemental

Outre que je ne trouve pas honteux d'avoir la prétention de changer le monde en s'appuyant sur l'émancipation humaine, permettez-moi de souligner que le dogmatisme dont vous faites preuve, et qui se veut moderne, ne cesse d'être contredit par les études internationales.

PME-TPE et grands groupes cotés en bourse, ni à la baisse du pouvoir d'achat de nos concitoyennes et concitoyens. En quoi est-ce ringard, en 2017, à l'heure du bond prodigieux des nouvelles technologies, de la révolution numérique, de défendre une semaine de travail non pas de 40 heures, ni même de 35 heures, mais de 32 heures, sans perte de salaire En quoi est-ce ringard de défendre le droit au repos et aux loisirs ? En quoi est-ce ringard de s'opposer aux licenciements motivés uniquement par l'augmentation des profits de quelques actionnaires déjà fort nantis ? Je ne peux m'empêcher de penser ici

pour les particuliers une fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG. On détourne l'attention de nos concitoyennes et de nos concitoyens, mais c'est là en réalité un coup terrible porté à la protection sociale

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, comme l'a souligné M. le rapporteur, le présent projet de loi retient un grand nombre de propositions qui ont déjà été défendues par le Sénat. Depuis longtemps, en effet, nous dénonçons le décalage existant entre la réalité des relations de travail et le cadre légal dans lequel vivent les entreprises et les salariés français. Nous avons plaidé pour la primauté de l'accord d'entreprise, que nous retrouvons dans le présent texte, en partant du principe que la prise de décision doit se faire au plus près des acteurs, là où la relation de travail s'établit et où les objectifs de l'entreprise sont réalisés. Nous avons demandé la réduction de la durée des procédures judiciaires, qui est tout de même, en moyenne, de vingt et un mois en France ! Nous avons recommandé la fusion des instances représentatives du personnel, pour simplifier les prises de décision, et expliqué l'utilité des contrats de mission. Nous avons à plusieurs reprises déploré l'incroyable complexité des formalités imposées aux employeurs par la création du compte de prévention de la pénibilité. Par une ironie des destins politiques, le présent projet de loi prévoit des dispositions inscrites dans un premier temps dans le projet de loi « travail », puis abandonnées sous la pression des syndicats et des « frondeurs ». Ce fut le cas, notamment, de la création d'un barème obligatoire harmonisant les dommages et intérêts versés au salarié en cas de licenciement abusif. La France est l'un des rares pays à ne pas prévoir de plafond pour ces indemnités, et leur montant peut varier du simple au triple ! Cela crée une grande insécurité juridique pour les employeurs, notamment les TPE-PME, qui voudraient embaucher.

de longues discussions, la défense d'un périmètre national permettant d'apprécier les difficultés d'une filiale d'un groupe licenciant en France. De nouveau, la sécurisation des règles du licenciement était oubliée, l'on maintenait des règles plus restrictives que celles qui existent dans la majorité des autres pays européens. Dès lors, comment s'étonner que les investisseurs fuient notre pays et son cortège de rigidités ? Le présent projet de loi tendrait à revenir sur ces tentatives avortées du précédent gouvernement. J'emploie le conditionnel car, malheureusement, si nous connaissons la plupart des intentions du Gouvernement, grâce aux déclarations qui ont accompagné sa communication,

Tout d'abord, le flou entoure la plupart des articles. Vous nous répondrez, madame la ministre, que les précisions figureront dans les ordonnances. Mais un projet de loi d'habilitation, s'il fixe des objectifs, doit également indiquer le positionnement qui leur est attaché. Or, ici, même sur des sujets très importants, nous ne pouvons avoir aucune certitude, en raison du parallélisme entre l'examen du texte par le Parlement et la tenue de négociations avec les partenaires sociaux. Le travail parlementaire s'en trouve faussé. trouve faussé. Par exemple, à l'article 1, un sujet important est évoqué, celui de la qualification du licenciement d'un salarié ayant refusé une modification de son contrat de travail par un accord de flexisécurité. Le texte du projet de loi vise simplement « l'harmonisation du régime juridique de la rupture du contrat de travail Or, de la nature d'un tel licenciement dépendra concrètement l'instauration ou non d'un plan de sauvegarde de l'emploi par l'entreprise, procédure lourde et contraignante. Vos déclarations sur le sujet, madame la ministre, traduisent votre volonté d'éviter une telle procédure, mais que sortira-t-il du texte issu de la concertation ? Nous savons qu'il s'agit d'un point de friction majeur avec les syndicats.

permettre à un employeur de prendre l'initiative d'un référendum lorsqu'il n'a pas été possible d'obtenir un accord majoritaire. Toutefois, la neutralité du texte permet n'importe quelle interprétation. Si le projet de loi n'apporte pas plus de précisions, si l'étude d'impact ne remplit pas son rôle, le texte devient une coquille vide, et l'accord des parlementaires reposera sur du sable. Rien n'est tranché, tout est remis aux « aléas » de la concertation. Vous me direz que nous aurons l'occasion de voter une seconde fois, sur le projet de loi de ratification des ordonnances, mais tout sera déjà joué en réalité, puisque les ordonnances entreront en vigueur dès leur publication au, notre vote leur permettant simplement d'acquérir force de loi.

Notre groupe, partageant le même esprit constructif, a déposé des amendements de simplification, afin de régler certaines difficultés rencontrées au quotidien par les entreprises. Ce projet de loi fait figure de test, car si les concessions devaient s'y développer, il pourrait finir par ne plus ressembler du tout à ce qui était annoncé. Nous ne pouvons que vous alerter, madame la ministre, sur la désillusion que constituerait, pour les entrepreneurs, une loi qui ne déverrouillerait rien et qui complexifierait au et qui complexifierait au lieu de simplifier. Je forme donc le voeu que les précisions apportées par le Sénat soient validées par le Gouvernement. Il s'agira ensuite d'aller plus loin. Le facteur déterminant d'une décision d'embauche reste l'activité, le carnet de commandes. Les emplois sont créés s'il existe une dynamique économique dans le pays et si les entreprises peuvent s'y développer. La Banque de France vient de relever sa prévision de croissance pour la France à 1,6 % en 2017, en raison d'une amélioration de l'environnement européen. C'est une reprise, mais elle reste modérée. Je rappelle que la France se situe en dessous des 2 % de croissance de la zone euro. Pour aller au-delà, il faudra davantage qu'un assouplissement de la réglementation sociale ; il faudra d'importantes réformes structurelles. là d'un autre débat, que nous devrons avoir le plus rapidement possible, dans le respect du pouvoir d'initiative et de contrôle des parlementaires. Notre vote sur ce texte représentera une première étape

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les Français, aujourd'hui trop nombreux à être écartés du marché du travail, demandent que nous oeuvrions à l'émergence de solutions pour enrayer ce terrible fléau qu'est le chômage. Si je partage le diagnostic établi par le Gouvernement d'un monde du travail entré dans une phase de profonds changements du fait de la mondialisation de l'économie, de la transition écologique ou de la révolution numérique, je suis en désaccord avec la méthode adoptée. Je note aussi des oublis, rien n'étant prévu, par exemple, en matière de médecine du travail. J'avais espéré, madame la ministre, que votre ambition était d'ajuster notre modèle social et d'affronter les mutations qui sont déjà à l'oeuvre. Or, dans ce texte, je ne vois pas la « flexisécurité à la française » tant promise ! Ce constat est encore aggravé par le démantèlement du code du travail opéré par la droite sénatoriale majoritaire, qui profite de ce projet de loi pour rogner sur les droits des salariés et rendre notre marché du travail toujours plus précaire,

d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale, qui précisait le champ du présent projet de loi d'habilitation et des futures ordonnances en y intégrant l'objectif d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l'entreprise. Ce n'est pas acceptable Je souhaiterais revenir, tout d'abord, sur la méthode. Très récemment, à Versailles, le Président de la République insistait sur sa volonté de revaloriser le rôle du Parlement pour légiférer mieux, dans la concertation. Je partage totalement ce point de vue. Si je ne suis évidemment pas opposée au principe du recours aux ordonnances, tel que prévu par l'article 38 de notre Constitution, je regrette que le Gouvernement agisse aujourd'hui dans la précipitation. La concertation sociale n'est pas encore terminée que nous sommes amenés à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances. En somme, vous nous demandez de vous autoriser à oeuvrer à notre place et en notre nom pour refondre entièrement le code du travail et notre modèle social ! Au moment où nous examinons ce projet de loi d'habilitation, il nous est encore impossible d'apprécier avec justesse l'équilibre de la réforme, entre la sécurité que vous promettez et la flexibilité que vous nous proposez. le recours aux ordonnances a pu se justifier par le passé, lorsqu'il s'est agi de mettre en oeuvre un véritable progrès social avec la cinquième semaine de congés payés ou la retraite à 60 ans, rien ne justifie aujourd'hui un tel empressement pour rendre les règles de licenciement plus souples, développer les CDI dits « de chantier », plafonner les indemnités de licenciement prud'homales, fusionner les instances représentatives du personnel ou faire évoluer le compte pénibilité.

Ne pouvait-on pas faire une évaluation des réformes passées, notamment la loi de Mme El Khomri ou la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, avant de s'orienter vers une refonte de notre droit du travail ? ? Un examen du détail des dispositions qui nous sont soumises montre que ni l'urgence, ni la portée, ni la technicité des sujets ne justifiaient, en fin de compte, ce recours aux ordonnances. de la méthode, je m'inquiète aussi du contenu de l'article 5, visant à reformer le compte personnel de prévention de la pénibilité, le C3P. Avec ce texte, le C3P est transformé en simple compte personnel de prévention.

partir plus tôt à la retraite, se former ou travailler à temps partiel sans perte de salaire. Si certains critères ne posent pas de problème, comme celui du travail répétitif ou de nuit, le Gouvernement souhaite écarter du dispositif quatre critères d'une importance majeure : la manutention manuelle des charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les risques chimiques. Pour ces quatre critères, on ne sera plus dans une logique de prévention : il s'agira uniquement de permettre à ceux qui sont atteints d'une invalidité de plus de 10 % de partir à la retraite plus tôt.

Pourtant, dans son discours de politique générale, le Premier ministre avait déclaré que la prévention serait le pivot de la stratégie nationale de santé devant être examinée à l'automne. à l'automne. Dans les faits, les entreprises ne seront plus véritablement incitées à réduire les situations de travail pénible. À cet instant, mes pensées vont aux salariés de l'entreprise Tréfimétaux de Dives-sur-Mer, dans mon département du Calvados, ainsi qu'à ceux de la « vallée de la mort », près de Condé-sur-Noireau, malades de l'amiante, qui a déjà causé bien trop de décès. Cet exemple de l'amiante illustre parfaitement l'impossibilité de réparer des maladies professionnelles qui se déclarent après le départ à la retraite. On nous dit que le dispositif serait trop complexe, qu'il engendrerait trop de bureaucratie pour les PME. Je veux bien l'entendre, mais je note tout de même que certaines branches

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je tiens, dans un premier temps, à saluer l'engagement du Gouvernement, dont l'un des premiers actes est d'entreprendre la réforme du dialogue social, nécessaire au développement de l'emploi en France. Je tiens également à féliciter notre rapporteur, Alain Milon, pour la qualité de ses travaux, sa mobilisation dans des délais extrêmement courts et la pertinence de son rapport. Nos échanges avec l'ensemble des partenaires sociaux, en commission, ont été riches d'enseignements. Nous entamons l'examen du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, texte qui introduira la première d'une longue série de réformes sociales annoncées par le Gouvernement. En effet, tous les acteurs économiques et la grande majorité des partenaires sociaux s'accordent à dire qu'une plus grande souplesse du code du travail et le développement d'outils de dialogue dans l'entreprise peuvent permettre de sécuriser à la fois les salariés dans leur parcours professionnel et les entreprises dans leur phase de développement. Même si cette simplification ne constituera pas, à elle seule, la réponse dans le combat collectif que nous devons mener contre le chômage, elle est un des atouts nécessaires à la relance économique et sociale que nous attendons tous.

Je tiens à souligner que je partage le sentiment de notre rapporteur quant à la méthode employée par le Gouvernement. Je peux comprendre que, eu égard à la situation économique de notre pays, le temps presse et qu'il faille aller vite, mais le fait de légiférer sur l'habilitation alors même que les négociations entre le Gouvernement et les partenaires sociaux sont en cours ne nous permet pas d'appréhender avec sérénité tous les enjeux dans le calendrier donné. Le texte que nous allons voter doit permettre de moderniser le dialogue social dans l'ensemble des entreprises, notamment en prenant en considération les particularités des PME et des TPE. Nous disposons d'un vivier de petites entreprises, innovantes, imaginatives, combatives, qui se débattent au quotidien pour gagner des marchés, trouver du personnel compétent et motivé, s'adapter aux nouveaux besoins et faire face à la concurrence. Rappelons que, en France, 95 % des entreprises sont des TPE et des PME de moins de cinquante salariés, et que 55 % de l'emploi salarié se situe dans ces entreprises. Ce sont elles qui créent des emplois et peuvent en créer plus encore.

dépourvues de délégué syndical, de conclure des accords collectifs directement avec les représentants du personnel ou, en leur absence, avec le personnel ». La commission des affaires sociales a également tenu à permettre à l'employeur d'organiser une consultation des salariés pour valider un accord. J'ai souhaité aller plus loin, en déposant un amendement tendant à permettre à l'employeur, dans les entreprises employant moins de onze salariés et dans les entreprises employant moins de cinquante salariés dépourvues de représentant du personnel, d'appliquer un accord type ou de prendre une décision unilatérale dans les domaines et les conditions prévus dans l'accord de branche.

Je m'attacherai aussi à la proposition d'étendre le contrat de chantier à d'autres secteurs que le bâtiment. Il s'agit, là encore, de se donner de la souplesse. Rappelons qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée par lequel un employeur engage un salarié pour la réalisation d'un ouvrage, de travaux ou d'opérations précis, mais dont la durée ne peut être préalablement définie avec certitude. Le salarié bénéficiera de davantage de visibilité que s'il enchaîne des CDD ou des contrats d'intérim.

Pour aller plus loin, je soutiens l'idée de créer un contrat de croissance. Une entreprise confrontée à une croissance soudaine à la suite de la conclusion d'un nouveau marché qui lui apporte un surcroît de travail sur plusieurs mois, voire plusieurs années, pourrait conclure ce type de CDI afin de s'adjoindre les compétences dont elle a besoin.

la loi. Afin de sécuriser les plus petites entreprises et les artisans qui ne sont pas dotés de service juridique, la commission a adopté, à l'article 3, un amendement tendant à permettre à l'employeur de « rectifier dans la lettre de licenciement les irrégularités de motivation si elles sont sans incidence sur la cause réelle et sérieuse du licenciement ». Cet amendement introduit dans notre législation l'ébauche d'un droit à l'erreur, attendu par les PME et les TPE. Il est temps de créer ce droit à l'erreur pour les chefs de petite entreprise, souvent de bonne foi, qui se voient suspectés, sanctionnés pour une simple erreur matérielle. Je salue également l'initiative du Premier ministre, qui a enfin proposé de simplifier le C3P, source de tracasseries administratives, véritable usine à gaz pour les entreprises, et de mettre en place un compte professionnel de prévention. À titre personnel, j'aurais préféré la suppression pure et simple de ce compte et la mise en place de mesures générales pour prendre en considération la pénibilité.

mais les chefs d'entreprise ont surtout besoin de conseils, d'accompagnement, que ce soit pour leurs projets de développement ou en période de difficultés. Une relation de confiance doit être développée, encouragée. Elle sera elle-même source de croissance et de création d'emplois.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président-rapporteur, la discussion que nous menons aujourd'hui est évidemment source de frustration pour les parlementaires que nous sommes. Nous travaillons sur un texte d'habilitation portant sur des mesures dont nous ne connaissons pas la teneur précise, les discussions avec les syndicats venant de s'achever et la rédaction des ordonnances n'ayant pas commencé. Le Gouvernement a choisi d'oeuvrer dans l'urgence, sans nous mettre réellement à contribution. Pour autant, cela n'est en rien une surprise : le Président de la République avait annoncé ses intentions lors de la campagne, et les ordonnances sont un moyen constitutionnel de légiférer.

bien sûr, des réserves. Nous partageons en partie le diagnostic : la situation du marché du travail n'est pas satisfaisante et il faut y remédier. Le rôle social du travail est essentiel et la lutte contre le chômage doit demeurer le coeur de nos priorités. Nous sommes nombreux à être favorables à une refonte du droit du travail, afin de mieux l'adapter aux bouleversements liés, notamment, aux nouvelles technologies et au numérique. Nous sortons toutefois d'un quinquennat riche en réformes dans ce domaine.

Je tiens par ailleurs à souligner que les réformes menées par la précédente majorité commencent à porter leurs fruits. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'ACOSS, a récemment annoncé que 2 millions d'embauches ont été déclarées au deuxième trimestre de 2017, dont près de la moitié en CDI. Le dispositif « embauche PME » n'y est sans doute pas pour rien ! Il convient de s'interroger sur l'opportunité d'accumuler les réformes avant de connaître les effets réels de celles qui ont déjà été engagées. Je demande donc au nouveau gouvernement et à vous-même, madame la ministre, d'être intransigeants sur l'évaluation des dispositifs mis en place. Le texte que nous étudions aujourd'hui vise seulement à déterminer le champ d'intervention des ordonnances à venir. Il est donc bien compliqué d'avoir un débat sur le fond, alors même que les négociations avec les organisations syndicales viennent de s'achever. Nous reconnaissons d'ailleurs la réalité du dialogue mis en place, que nous saluons. Nous demandons simplement, madame la ministre, que vous soyez extrêmement attentive aux revendications des syndicats de salariés. En effet, nous souhaitons que vous aboutissiez à des textes équilibrés. Il est indispensable de renforcer les garanties accordées aux salariés et aux travailleurs indépendants. Sécuriser les employeurs ? D'accord, si cela peut favoriser les embauches, mais il doit y avoir des contreparties en termes de bien-être des salariés. Nous serons donc particulièrement vigilants au moment d'examiner le contenu des ordonnances, s'agissant notamment du travail de nuit, qui doit rester exceptionnel. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale nous rappelle régulièrement, dans ses rapports, que le travail de nuit comporte des risques pour la santé. Il doit donc être particulièrement encadré. Nous serons également prudents en ce qui concerne le champ du CDI de chantier. Pourquoi ne pas l'étendre à des missions précises, dès lors qu'elles sont limitées dans le temps, si cela peut favoriser l'embauche ? Cependant, ce type de contrat ne doit en aucun cas devenir la norme. Son utilisation doit rester circonscrite à des domaines spécifiques et clairement identifiés. Nous serons aussi attentifs à l'éventuelle mise en place d'un barème obligatoire pour le calcul des indemnités prud'homales en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les syndicats de magistrats s'en inquiètent selon eux, elle empiéterait sur le pouvoir d'appréciation des juges et déséquilibrerait le rapport de force entre employeurs et salariés. Par ailleurs, la réforme votée en 2015 créant un barème indicatif commence juste à entrer en vigueur pourquoi ne pas procéder à une évaluation de cette mesure avant de se précipiter pour mettre en place un barème impératif ? Enfin, nous sommes très attachés au compte personnel de prévention de la pénibilité.

Ils ont explicitement ouvert la voie, à l'alinéa 13 de l'article 1, au référendum d'entreprise sur l'initiative de l'employeur. Cela permettrait à ce dernier de court-circuiter les organisations représentatives du personnel et lui conférerait une marge de manoeuvre bien trop importante, compte tenu de la relation de subordination existant entre lui et les salariés. Les modifications apportées à l'article 3 ne nous conviennent guère plus. Nous ne souhaitons pas la réduction de moitié du délai de contestation d'un licenciement économique, qui est aujourd'hui d'un an. de la possibilité, pour les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégué syndical, de « conclure des accords collectifs directement avec les représentants élus du personnel ». Accorder un droit à l'erreur à l'employeur en matière de rédaction des lettres de licenciement ne nous paraît pas non plus nécessaire. Nous ne souscrivons pas davantage, à ce stade de la procédure législative, à la limitation à trois du nombre de mandats consécutifs pour les membres de la future « instance unique » de représentation des salariés. Mes chers collègues, nous devrons patienter jusqu'à la discussion des textes de ratification des ordonnances pour débattre sur le fond. C'est à ce moment-là seulement que nous pourrons examiner des mesures concrètes. En attendant, nous considérons que le texte adopté par la commission des affaires sociales du Sénat a été déséquilibré par la majorité sénatoriale : elle a donné au cadre que constitue cette loi d'habilitation la forme d'un trapèze penchant vers les intérêts du patronat et la flexibilité sans restriction. Nous nous y opposons.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président-rapporteur, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner le projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

: des délais très contraints, une concertation avec les partenaires sociaux qui n'est pas terminée et le recours aux ordonnances, couvrant un champ immense. Pour autant, Pour autant, en tant que membre de la délégation sénatoriale aux entreprises, je me réjouis de l'orientation générale de ce texte, car nos entreprises devraient pouvoir gagner en simplification, et donc en compétitivité. L'emploi devrait, par voie de conséquence, en bénéficier.

À cette surréglementation s'ajoutent l'instabilité du droit et l'insécurité juridique permanente due à la prolifération de règlements complexes, non différenciés en fonction de la taille de l'entreprise. ces conditions, si les objectifs du Gouvernement sont de redonner du sens au dialogue social, de rationaliser les institutions représentatives du personnel, de libérer l'embauche, nous ne pouvons que nous en féliciter Pour autant, si notre ambition est de promouvoir une société du travail, d'instaurer un climat de confiance avec les chefs d'entreprise pour créer des conditions favorables à l'embauche, nous devons aller plus loin.

simplifie le droit du travail, au profit des salariés et des employeurs. Il faut dire que la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a encore complexifié la législation, notamment pour les TPE-PME. Le droit actuel ne leur permet pas de s'adapter à la réalité des situations économiques, par exemple en zone de montagne, où elle se caractérise par le recours à l'emploi saisonnier. L'article 1 doit permettre de sauvegarder le rôle essentiel de la branche professionnelle et de conclure des accords collectifs directement avec les représentants du personnel.

à la simplification des instances de représentation du personnel, avec la mise en place d'une instance unique, compétente en matière de négociation des accords d'entreprise. Bien sûr, la sécurisation juridique des procédures de licenciement doit être mieux appréciée et les délais de contestation, comme les critères d'appréciation, doivent être davantage précisés à l'article 3. S'agissant du compte personnel de prévention de la pénibilité, sa mise en oeuvre sur le terrain a été un véritable échec et je suis favorable à sa transformation, comme proposé à l'article 5, en compte personnel de prévention, moins contraignant pour l'employeur, mais tout aussi favorable à l'employé. Je voudrais m'exprimer plus en détail sur l'article 9, qui vise à reporter au 1 janvier 2019 le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. En effet, même si ce report est déjà une bonne chose, qu'il me soit permis de vous sensibiliser sur l'impact d'une telle mesure pour les entreprises. Le 28 juin dernier, dans le cadre de la délégation sénatoriale aux entreprises, une étude d'impact réalisée par le cabinet Taj nous a été présentée. Outre la complexité des mécanismes du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, deux aspects importants ont été relevés : le coût que représente cette mesure pour les entreprises et le ressenti des employés et des employeurs. Le coût administratif de la collecte, supporté par les seules entreprises, a été estimé à 1,2 milliard d'euros l'année de la mise en place Quant au coût récurrent, il est évalué à 100 millions d'euros par an. Cette réforme touchera en priorité les TPE, à hauteur de 70 %, puisqu'elles sont aujourd'hui en France au nombre La réforme prévoit que les très petites entreprises, comptant moins de 10 salariés, pourront conserver pendant trois mois l'impôt dans leur trésorerie. Or cette mesure ne représente aucun gain financier pour les entreprises, eu égard au taux d'intérêt bancaire moyen. Je me réjouis donc de l'adoption d'un amendement de notre collègue Albéric de Montgolfier instituant un prélèvement contemporain de l'impôt, fondé sur la transmission instantanée par les entreprises des informations sur les salaires, ce prélèvement étant effectué non plus par les entreprises, mais bien par l'administration fiscale. En ce qui concerne les effets psychologiques de cette mesure, ils sont bien réels, même s'ils sont difficilement quantifiables, et leur impact pourrait dégrader le climat social au sein des entreprises, le salarié pouvant légitimement considérer que son employeur s'immisce dans sa vie privée. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, ce texte est loin d'être neutre. Il implique des changements importants en termes de rénovation de notre modèle social, des changements profonds du côté tant des employeurs que des employés. Pour échanger régulièrement avec les uns comme avec les autres, je sais que l'ensemble des acteurs, sur le terrain, sont prêts à se saisir de ces nouvelles opportunités. Pour toutes ces raisons, je suis plutôt favorable à ce projet de loi, mais je serai très attentive aux différents amendements qui seront examinés en séance publique.

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues,

les syndicats, sous prétexte de défendre les salariés, ne se préoccupent jamais de l'avenir des entreprises. Certaines ont fait faillite faute d'avoir pu licencier le personnel surabondant qu'elles ne pouvaient plus payer. Les salariés ont intérêt

Il faudra bien expliquer à l'opinion et aux salariés que la précarité est le fondement même de l'emploi. Rien n'est éternel : la vie, la santé, les mandats électoraux et l'emploi sont précaires. Seuls les emplois de fonctionnaire ne le sont pas, mais ils sont payés par l'État, qui a des moyens que les entreprises n'ont pas. Que les syndicats cessent de croire

leur activité. Madame la ministre, j'espère que vous pourrez convaincre, par une large campagne d'information, tous les salariés et les jeunes de ne pas suivre les éventuelles consignes de grève des syndicats, car cela les conduirait au chômage.

Permettez-moi de retracer brièvement mon expérience personnelle dans ce domaine. Quand j'ai pris le contrôle de Dassault Aviation, en 1986, il n'y avait pas assez de commandes et les caisses étaient vides. J'ai réuni le personnel- et pas les syndicats -et lui ai dit que, pour préparer l'avenir, il fallait que je dispose de moyens suffisants pour étudier et construire de nouveaux prototypes. Dans cette perspective, je leur ai

Au bout de trois ans, j'ai mis en place un accord de participation dérogatoire qui a permis que, après autofinancement, le bénéfice distribuable soit divisé en deux parts égales : une pour les actionnaires, l'autre pour les salariés.

Ce qui est bien dans votre système, c'est que nous ne travaillons plus uniquement pour le patron, mais aussi pour nous.

de dernier message, permettez-moi de vous rappeler qu'il faut tout faire pour annuler nos divisions gauche-droite, qui nuisent à notre développement économique et à notre paix sociale. Elles n'existent plus dans de nombreux pays et elles ne mènent à rien. N'oubliez pas, mes chers collègues, qu'il n'y a pas un peuple de gauche et un peuple de droite, mais un peuple de France, qui doit pouvoir travailler pour le bien de tous. Le président Emmanuel Macron a dit qu'il n'était ni de gauche ni de droite ; il a raison, c'est la bonne voie.